dans ces périodes de désarroi, chacun peut comprendre les souffrances exprimées. La crise que traverse notre pays depuis l'automne dernier montre les fractures auxquelles le Gouvernement, les élus nationaux et les élus locaux doivent répondre : fracture sociale et fracture territoriale, mais aussi crise de confiance. Face au malaise exprimé par nos concitoyens, chacun essaie de mieux écouter. C'est ce que nous faisons tous actuellement

rien ne justifie les provocations contre la République. Quand plus aucun symbole n'est respecté, comment s'étonner de la résurgence de comportements que nous pensions définitivement appartenir au passé ? La nausée que nous inspire la résurgence de l'antisémitisme, tout comme les récentes profanations d'églises, renforce notre détermination à ne jamais rien céder quand l'essentiel est en jeu. Un certain nombre d'élus- députés, sénateurs, élus locaux -ont récemment été victimes d'agressions ou de menaces. Certains ont vu leurs locaux vandalisés. Je veux locaux vandalisés. Je veux exprimer ici la solidarité du Sénat à leur égard et adresser un message de soutien tout particulier au président de l'Assemblée nationale, notre collègue Richard Ferrand. Attaquer des hommes et des femmes qui investissent une grande partie de leur vie dans la défense de l'intérêt général et qui s'engagent au service de leurs concitoyens, c'est nier la démocratie, c'est malmener la République. L'ordre du jour appelle les

L'ordre du jour appelle les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public solennel sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Merci

les termes du rapport Notat. Trois mois de débats préparatoires, un mois de débats en ligne, une discussion approfondie en commission spéciale à l'Assemblée nationale

la création d'une procédure d'opposition aux brevets, ou encore à la représentation plus équilibrée des femmes dans les fonctions exécutives des sociétés.

suppression de l'interdiction de la fabrication de certains produits phytopharmaceutiques, l'autorisation, sous conditions, de l'ouverture des commerces de détail alimentaire le dimanche après-midi,

ADP, le Sénat a rayé d'un trait de plume toutes les améliorations que le rapporteur avait apportées au dispositif adopté par l'Assemblée nationale : cahier des charges, conditions de la régulation, surveillance des différents tarifs.

Pour notre part, nous sommes heureux qu'une majorité d'idées se soit dégagée pour refuser la privatisation et le bradage du monopole naturel que constitue ADP.

celui de l'aéroport de Toulouse-Blagnac et celui à venir de nos barrages hydroélectriques, voilà un premier coup d'arrêt dans la vente de nos actifs dans des secteurs stratégiques de l'État.

Quant à vous, monsieur le ministre, il vous faudra respecter la voix du Sénat. Il est inconcevable, dans le moment politique que nous traversons, que vous puissiez passer outre cette quasi-unanimité. Envoyer un message Envoyer un message contraire serait désastreux, au moment où vous prônez le dialogue partout dans le pays. Nous vous faisons une proposition : sortez de ce projet de loi les privatisations et intégrez cette question dans le grand débat national. Êtes-vous d'accord

Pour le reste du texte, il y a un fil rouge cohérent : amplifier, sous couvert de vouloir « moderniser et simplifier », le détricotage du code du travail. En réalité, vous voulez créer un nouveau western social, où la loi du plus fort deviendra la norme. Par exemple, en deux cents articles, il n'y a aucun droit nouveau pour les salariés L'entreprise serait au coeur de votre projet de loi, mais pas les entrepreneurs, ni les salariés, ni les sous-traitants, ni les collectivités territoriales ! Comment comprendre qu'un certain nombre de nos amendements répondant à l'intérêt général, faisant écho à la crise sociale que nous traversons et en lien avec le texte aient été déclarés irrecevables ou refusés ? Augmenter le SMIC ? Pas à l'ordre du jour ! Augmenter les salaires

Vous n'y pensez pas, nous ne sommes pas en Union soviétique ! » C'est vrai ! Au terme de cette discussion, on ne sait plus,, si ce texte sert l'intérêt général ou des intérêts particuliers ! Comment comprendre que nous ayons passé près de deux heures de débat pour renforcer la place de Paris au bénéfice de quelques centaines de traders londoniens qui seraient tentés de venir chez nous en raison du Brexit, alors que nous n'avons, à aucun moment, traité de la question de la relation entre donneurs d'ordres

financiarisation accrue des entreprises, renforcement du secret des affaires l'opacité des comptes, attaques contre nos mécanismes nationaux de solidarité et fragilisation des droits des salariés, changements de gouvernance pour la Caisse des dépôts et consignations et La Poste, ou encore casse des seuils sociaux. sociaux. Le Medef en rêvait, la droite ne l'avait pas fait, vous l'avez enfin réalisé ! Mettre à bas les seuils sociaux ! Cette mesure devrait autant participer à la création emploi que le CICE, c'est-à-dire à un Mais vous avez réussi à faire croire que la présence syndicale, la représentation des salariés, un certain nombre de droits qui leur seraient concédés constitueraient un frein au dynamisme de nos entreprises et à l'emploi. C'est d'autant plus dogmatique que, en 2017, les 47 % d'entreprises interrogées par l'INSEE déclarant rencontrer des « barrières à l'embauche » les associaient davantage à l'incertitude sur la situation économique et à la difficulté de trouver une main-d'oeuvre qualifiée qu'à la suppression des seuils sociaux. Un jour, monsieur le ministre, il faudra nous dire quelle est votre vision de la société. Une société où il n'y a en fait qu'une seule

obligations, des règles, des contraintes, dont les entreprises devraient être libérées, car elles empêcheraient l'embauche dans notre pays. Pourtant, nous devrions être fiers de notre modèle social et le défendre plutôt que tout faire pour le tuer à petit feu. Le monde entier nous l'envie ! Les cotisations sociales permettent de remplir les caisses de la sécurité sociale, et nous savons bien qu'un salarié bien soigné et bénéficiant d'une protection sociale est un salarié compétitif. Enfin, sur nombre d'articles, votre texte tombe à plat. Vous parlez d'intéressement et de participation sans parler de partage de richesses ni de salaires. Nous avons travaillé sur une légère refonte de l'épargne retraite, alors que, en ce moment même, M. Delevoye conduit une consultation pour mettre à bas notre système par répartition. Vous évoquez le statut d'auto-entrepreneur sans, à aucun moment, mentionner le fait que ce statut est dévoyé par des plateformes comme Uber ou Deliveroo pour exploiter des jeunes sans protection sociale. Heureusement que, parfois, les tribunaux vont plus vite que le législateur pour considérer que ces jeunes sont des salariés à part entière. Votre texte, monsieur le ministre, connaîtra le même sort que les cinq derniers qui étaient relatifs aux entreprises : il ne résoudra rien ! Au contraire, il aurait fallu écouter le murmure qui monte dans le pays : « Partagez le gâteau ! » Quel gâteau ? Et la cerise ? ... Je ne sais pas si c'est pour demain ou pour après-demain, mais ce jour arrive à grands pas. Les peuples en ont assez de souffrir pendant que d'autres accumulent des richesses. Alors, continuez à ne pas voir que ce système libéral s'écroule sous vos yeux et que l'espoir est revenu ! Comme le dit le poète Gibran Khalil Gibran, « les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés le matin à la table des anges

encore faut-il clairement identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans notre système. Et c'est peut-être là que le bât blesse Dans ce débat, le Sénat a eu un rôle essentiel : supprimer les privatisations d'ADP et de La

que la gauche et la droite défendent ensemble l'intérêt national, lorsqu'il s'agit de pépites publiques comme ces deux

On ne vend pas des bijoux de famille à des intérêts privés. Ces privatisations sont une aberration économique et une erreur politique.

de l'aéroport de Toulouse et à l'abandon de notre industrie. En privatisant ses entreprises, la France perd la maitrise de son destin et de ses moyens d'action. Monsieur le ministre, nous pensons que ce projet de loi PACTE est une occasion manquée.

contre l'économie sociale et solidaire, qui est symptomatique du caractère néolibéral de ce projet de loi. À l'heure où la sauvegarde de notre planète est devenue une priorité, les insuffisances de ce texte quant à l'environnement et au développement durable sont tout à fait incompréhensibles.

Vous avez refusé de limiter les hauts salaires, qui sont un vrai scandale, mettent à mal notre cohésion sociale et renforcent le sentiment d'injustice. La désindustrialisation est toujours en marche,

au « Rendre sa grandeur à l'Amérique », il est plus que jamais nécessaire d'avoir un État stratège et une Europe capable de rivaliser avec ces deux continents.

entreprises stratégiques, en ramenant à 10 % du capital, contre 25 % auparavant, le seuil lui permettant de mettre à l'étude ou de bloquer des acquisitions étrangères dans des entreprises

nous avons une plus haute ambition pour nos entreprises et l'avenir économique de notre pays. Nous pensons que de nouvelles régulations doivent s'imposer, avec un État stratège omniprésent.

dans la discussion générale, j'avais fait part de l'accueil favorable de ce texte par le groupe du RDSE, avec, bien sûr, quelques réserves, et en espérant que des améliorations et des enrichissements puissent être apportés par notre assemblée. L'une des difficultés rencontrées portait sur le champ extrêmement large de ce texte, ce qui a pu nuire à l'identification d'une ligne directrice claire. À mon sens, la cession des participations publiques et la gouvernance des grands groupes publics comme la Caisse des dépôts et consignations et La Poste auraient pu faire l'objet d'un texte distinct ; cela aurait été plus clair et plus cohérent. Sur l'ensemble, on ne pouvait que se féliciter des objectifs annoncés de transformation économique avec plus de liberté, de simplicité et d'efficacité pour les entreprises et les entrepreneurs. Finalement, le texte qui nous est proposé aujourd'hui répond-il à ces objectifs et a-t-il été vraiment amélioré pendant ces deux semaines de débat ? Permettez-moi d'en douter. Si le Sénat, par le texte adopté par sa commission spéciale ou par la voie d'amendements, a apporté un certain nombre de précisions utiles et d'enrichissements pertinents, ceux-ci concernent principalement des aspects techniques et ne portent pas sur l'essentiel. Il est impossible de balayer l'ensemble des thèmes abordés. Je n'évoquerai donc que ceux qui ont le plus animé les débats. En premier lieu, la cession et la modification du régime juridique d'Aéroports de Paris,

La privatisation de La Française des jeux ayant été évacuée d'emblée par la commission spéciale, le Gouvernement devra se consoler avec la seule validation du retrait de l'État d'Engie.

En ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat, l'acceptation d'une seule structure régionale a été obtenue à la suite d'un débat quelque peu confus, et je ne suis pas certain que le vote ait vraiment reflété la position de la majorité des sénateurs présents ce soir-là. cette évolution, comme c'est le cas pour de nombreuses autres structures économiques, professionnelles, administratives, associatives, sportives ou culturelles, s'inscrit dans une tendance lourde de centralisation des pouvoirs et des moyens financiers C'est une conséquence de la loi NOTRe, même si le processus était déjà engagé auparavant. C'est une voie qui va continuer d'affaiblir les territoires périphériques, notamment ruraux, sans nécessairement gagner en efficacité. À mon sens, c'est tout l'inverse d'une politique de décentralisation et de proximité. Le troisième thème de ce texte, « Des entreprises plus justes », contient des mesures très positives concernant l'épargne salariale et l'actionnariat des salariés avec un apport significatif du Sénat. Je ne ferai que regretter le rejet d'un amendement visant à élargir le champ d'application de l'intéressement obligatoire à toutes les entreprises de plus de dix salariés. Je suis persuadé qu'un jour cette mesure s'imposera d'elle-même, mais le Gouvernement et le Sénat se refusent pour l'instant à aller plus vite dans ce domaine, sachant pourtant que la méthode incitative n'aura que des effets limités sur le nombre de salariés bénéficiaires de ce dispositif. Je suis prêt à prendre le pari qu'une telle mesure Enfin, dernier point chaud, si je puis m'exprimer ainsi, le relèvement du seuil de 50 à 100 salariés. C'était une mesure emblématique, apparemment séduisante pour les entreprises et à laquelle je pourrais souscrire. Même si ce n'est qu'un affichage, dont les auteurs savent qu'il n'a que peu de chances d'être retenu à l'Assemblée nationale, cette disposition contient quelques effets pervers qui, me semble-t-il, ont été sous-estimés. Cette mesure est finalement assez discutable, car elle se justifie moins du fait de la fusion des instances de représentation du personnel en une seule structure depuis les ordonnances Travail. En outre, elle risque de rendre plus difficile la définition de mesures spécifiques en faveur des petites entreprises et elle supprime la garantie pour tous les salariés des entreprises de 50 à 100 salariés de bénéficier de la participation c'est donc une régression en termes de partage des résultats. Je ne suis pas sûr que ceux qui ont voté cette mesure ne souhaitent pas aujourd'hui que l'Assemblée nationale ne nous suive pas sur ce point ... Parmi mes regrets, je pourrais encore citer le report de 2020 à 2021 de l'application du relèvement des seuils du contrôle légal des comptes des sociétés. Cette décision n'est pas compréhensible pour les entreprises, mais il convient de reconnaître que la profession de commissaire aux comptes est bien organisée.

comme je l'avais indiqué lors de la discussion générale, ce texte aurait gagné en cohérence, si son périmètre avait été mieux ajusté. Pour autant, il faut reconnaître que le travail de la commission spéciale et de la Haute Assemblée l'a amélioré sur de nombreux points, même si, à titre personnel, je regrette que des sujets importants n'aient pas été suffisamment pris en compte ou écartés à tort- j'y reviendrai Indiscutablement, le point fort de ce texte porte sur la modification des seuils. Je souhaite que le Gouvernement et l'Assemblée nationale ne reviennent pas sur les décisions que nous avons prises, car elles représentent, à elles seules, la bouffée d'oxygène réglementaire qu'attendent nos entreprises. La France et les Français iraient mieux si l'économie et l'emploi étaient plus performants. Ces mesures n'ont pas de coût budgétaire pour le Gouvernement, mais elles peuvent changer l'état d'esprit et les résultats de nos entreprises. Nous en avons grand besoin S'agissant des chambres consulaires, même si nous y avons apporté des modifications, je regrette que le texte final ne donne pas plus d'importance à la liberté d'organisation et à la responsabilisation des acteurs de terrain. Toutes ces nouvelles organisations vont, finalement, amener les chambres à facturer leurs services pour compenser les ponctions opérées sur leurs budgets, alors même qu'il n'y a aucune baisse ni suppression des taxes qui les alimentaient. Les entreprises paieront donc deux fois En ce qui concerne ADP et La Française des jeux, la suppression des privatisations me paraît être une bonne chose, car ces dossiers n'étaient pas suffisamment élaborés. Nous avons bien vu ce qu'a donné la privatisation mal maîtrisée des autoroutes. Je regrette que le Sénat ne m'ait pas suivi sur l'intérêt d'avoir un brevet de qualité face à nos voisins. Je pense que nous y reviendrons. La France n'a pas intérêt à être le réceptacle des brevets de faible intérêt, tandis que les bons brevets seraient pris ailleurs. Je regrette enfin que trop de nos propositions d'amendements se soient vues opposer une nouvelle lecture de l'article 45 et aient été L'obligation qui nous a été faite de ne partir que du texte initial du Gouvernement me paraît en contradiction avec la lettre de la Constitution, qui nous demande de partir du texte de la commission de l'Assemblée nationale. Cette méthode aura pour conséquence de priver le Sénat d'une capacité de peser sur les nouveautés apportées par les députés, donc de réduire notre poids, ce qui me paraît, à l'heure actuelle, de mauvaise politique. Monsieur le président, il nous faudra réexaminer l'application de l'article 45, qui met en danger notre assemblée. Voilà, mes chers collègues, des motifs de satisfaction et de regrets.

le groupe Union Centriste a abordé l'examen de ce texte avec enthousiasme, tant il est important que nous puissions soutenir le développement économique de notre pays. Nous avons entrepris de travailler sur ce texte dans cet esprit et, comme vient de le dire Philippe Adnot à l'instant,

voire quelques siècles. Il faut savoir évoluer avec son temps. Aujourd'hui, nous le savons, la prise en compte des aspects sociaux et environnementaux est absolument essentielle. Même le MEDEF va se doter d'une raison d'être.

nous nous apprêtons à voter le projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises. Je tiens tout d'abord, au nom du groupe Les Indépendants, à saluer à mon tour le travail mené par la commission spéciale, sous la présidence de notre collègue Catherine Fournier,

Ce vote va intervenir après une nouvelle vague d'agitation sociale. À ce sujet, monsieur le président, nous saluons votre condamnation extrêmement claire de toutes les violences et de tous les outrages, qui sont proprement inacceptables.

À la source de cette situation se trouvent en effet certains des problèmes que ce projet de loi se donne précisément l'ambition de résoudre. C'est le travail, qui ne paie pas assez, et ne permet plus toujours de vivre décemment. C'est l'administration, qui décourage inutilement les efforts accomplis. C'est le sentiment, enfin, que partagent nombre de nos concitoyens, d'être les perdants de la mondialisation. Le texte que nous nous apprêtons à voter redonnera du souffle à nos entreprises. C'est notre conviction. Il fera respirer notre économie en relâchant les carcans dans lesquels nous avons progressivement enfermé l'initiative individuelle. Nous pensons, enfin, qu'il contribuera utilement à restaurer la confiance dans la liberté d'entreprendre. La contribution du Sénat dans la construction de ce texte permet d'aller plus avant dans cette direction. Je pense notamment au relèvement des seuils de 50 salariés à 100 salariés, afin de donner à nos PME plus de temps pour répondre à leurs obligations légales. Cette disposition, couplée à la période de mise en conformité pour le franchissement des seuils, allégera fortement la pression normative qui contraint encore la croissance de nos PME. Le Sénat a aussi porté la voix des territoires dans ce débat. C'est notamment le sens d'un amendement que nous avons déposé avec d'autres collègues sur ces travées. Cet amendement visait à réintroduire la généralisation de l'organisation administrative du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat autour d'un établissement unique de région, tout en précisant les moyens d'action des chambres de niveau départemental. Il faut maintenir un réseau dense pour ces structures d'accompagnement, qui donnent accès à la création d'entreprise au coeur de nos territoires. Je me réjouis que le Sénat puisse ainsi se faire l'écho de ces voix des territoires. Elles nous alertent contre le risque d'une rupture toujours plus marquée entre les centres et les périphéries, entre la France qui trouve sa place dans la mondialisation et celle qui a l'impression d'y perdre. C'est notre rôle de veiller à ce que les lois n'ajoutent pas au sentiment d'abandon qui nourrit la frustration de tant de nos concitoyens. Il y va de la cohésion de notre société. Pourtant, mes chers collègues, nous devons également avoir conscience que, à l'issue de ces débats, la position du Sénat n'apparaîtra pas clairement sur certains sujets structurants, comme Michel Canevet l'a rappelé. En particulier, nous n'avons pas apporté de réponse univoque à une question essentielle qui nous était posée dans quelle mesure souhaitons-nous voir l'État intervenir dans notre économie ? Une majorité d'entre nous a ainsi refusé la privatisation de La Française des jeux, souhaité encadrer celle d'Aéroports de Paris et choisi de confirmer celle d'Engie. Sur le fond, ma position personnelle reste constante : ce qui relève du pouvoir régalien doit être géré par l'État ; le reste doit être délégué. Très bien ! Tout à fait ! J'ai du mal à voir, mes chers collègues, en quoi la gestion de l'énergie serait moins stratégique pour l'État que celle du tourisme ... Il

Au fond, il ne s'agit pas tant de savoir s'il nous appartient, à nous, législateurs, de décider si nous devons conserver ou non des actifs stratégiques pour l'État, que de déterminer si l'intervention de l'État se révèle stratégique pour ces actifs, dès lors que l'État ne faillit pas à l'exercice de ses missions régaliennes. Plus prosaïquement, je pense que nous remplirions mieux notre rôle en prenant une part active et constructive à la définition des modalités dans lesquelles les cessions d'actifs pourront s'opérer. J'ai déjà eu l'occasion de le dire alors que nous commencions l'examen de ce projet de loi : la transformation de notre économie ne se décrète pas ; ce sont les entreprises qui s'en chargeront elles-mêmes. Notre rôle doit d'abord consister à leur donner les outils les mieux adaptés aux évolutions de notre économie et en assurer un cadre juste. Nous devons laisser plus de liberté pour innover et inventer de nouvelles solutions aux problèmes de notre temps. À cet égard, je suis convaincu que des outils, tels que le statut d'entreprise à mission, dont le Sénat a tenu à clarifier et simplifier le régime, ainsi que la réduction du forfait social sur la participation et l'intéressement constituent des moyens concrets et efficaces de répondre à ces enjeux. Je suis certain que nos entreprises sauront s'en emparer pour façonner un modèle plus en phase avec les aspirations des Français, c'est-à-dire plus inclusif, plus juste et plus durable. C'est en nous efforçant de restaurer la confiance dans la société, plutôt qu'en créant de nouvelles barrières, que nous parviendrons, aujourd'hui et demain, à dynamiser la compétitivité de notre économie, tout en assurant la cohésion sociale. C'est le cas, aujourd'hui, avec la loi PACTE, et ce sera le cas, demain, avec d'autres projets de loi que nous aurons à examiner et qui se révéleront également déterminants pour la France. Nous devrons alors miser de nouveau sur la confiance, pour accélérer la transformation de notre société.

madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, au terme de l'examen de ce texte, je tiens tout d'abord à saluer la qualité du travail de la commission spéciale, de sa présidente et de ses trois rapporteurs. Ce texte est présenté par le Gouvernement comme le grand texte économique de ce quinquennat, paré d'un titre et de chapitres ambitieux : « Des entreprises libérées, plus innovantes, plus justes » ... Pour un peu, on chanterait. l'extrême diversité des sujets traités dans ce texte et leur inégale importance ne dégage pas, nous semble-t-il, le souffle nécessaire susceptible d'impulser le choc de compétitivité espéré par de nombreux chefs d'entreprise. Sur la forme, le texte est passé de 73 articles à près de 200 articles à l'issue de son examen à l'Assemblée nationale. Ainsi, nombre de dispositions, parfois sur des sujets majeurs, ont échappé à une véritable étude d'impact, l'exemple le plus flagrant étant cet amendement « anti-Huawei annoncé par voie de presse et déposé pour le moins tardivement par le Gouvernement, pendant l'examen même du texte. Sans nier l'importance du sujet, convenez qu'il était nécessaire d'expertiser sérieusement,, la solution proposée. Le Sénat l'a rejetée à regret, mais en toute responsabilité. Sur le fond, nous nous retrouvons, monsieur le ministre, sur le constat : les obstacles rencontrés par les entreprises, essentiellement les petites et les moyennes, pour se développer, créer des emplois, se sont sédimentées au fur et à mesure de l'évolution de la législation et de son adaptation aux nouveaux enjeux économiques. Bien des scories normatives entravent aujourd'hui une croissance agile et efficace des PME. Ce texte permet d'en simplifier un nombre certain. C'est dans cette perspective que les travaux du Sénat ont renforcé sensiblement le texte, tant en commission qu'en séance. En particulier, nous sommes allés plus loin sur la rationalisation des seuils, en relevant les obligations liées au passage de 50 salariés à 100 salariés. C'est le seuil le plus emblématique en matière de croissance des entreprises. Il serait souhaitable que la CMP puisse trouver un bon équilibre sur ce point, car c'est une mesure très attendue. Nous avons également rendu les dispositifs relatifs à l'épargne salariale encore plus attractifs, en alignant les taux dérogatoires du forfait social sur le taux de 10 tant pour le plan épargne retraite que pour la participation ou l'intéressement, des sujets auxquels le Sénat est particulièrement attaché. Nous nous félicitons de ces dispositions. En outre, nous avons renforcé le poids des élus dans le conseil d'administration de La Poste, en accompagnant sa transformation. Nous sommes allés plus loin pour sécuriser davantage le développement des levées de fonds en actifs numériques, avec une sanction pénale pour ceux qui tromperaient les épargnants. Enfin, nous avons permis une meilleure information et une meilleure protection des consommateurs dans le cadre de la fin des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. plusieurs sujets ont fait l'objet de désaccords entre le Gouvernement et notre Haute Assemblée, le Sénat ayant souhaité poser un regard différent sur le débat. Oui, nous avons supprimé la définition de l'intérêt social et de la raison d'être de l'entreprise dans le code civil : si nous partageons la volonté de voir nos entreprises se transformer et le souhait de les accompagner vers de nouveaux modèles de croissance plus sociaux, plus tournés vers les préoccupations environnementales, il nous est apparu que l'imprécision des termes de cet article allait fragiliser les entreprises et faire peser sur elles un risque de contentieux accru, alors que la législation française sur la responsabilité sociale D'ailleurs, certaines entreprises et organisations représentatives se sont d'ores et déjà dotées d'une raison d'être, en toute liberté, cher Michel Canevet, preuve, s'il en était besoin, qu'il n'y a pas besoin d'une loi pour le faire. Produit en Bretagne en est un bon exemple. La stratégie d'une entreprise, monsieur le ministre, est sa responsabilité, sa liberté, son ADN, et elle s'exprime dans son projet d'entreprise. Nous pensons que les lois doivent être normatives, plutôt que bavardes. Lorsque la loi ouvre de tels espaces d'interprétation, c'est la jurisprudence qui prend le pas sur le pouvoir politique. En ces temps de confusion institutionnelle, chacun doit être attentif à son rôle. Nous avons bien sûr, au terme de longs débats ayant mené à un quasi-consensus, renoncé aux privatisations d'Aéroport de Paris et de La Française des jeux. d'abord, la motivation présentée par le Gouvernement nous semblait peu convaincante : le rendement attendu du fonds de rupture est d'ores et déjà équivalent aux dividendes perçus par l'État au titre de ces sociétés. Nous comprenons que des dividendes peuvent naturellement fluctuer, mais admettez, d'une part, qu'il en va de même pour le rendement des fonds de placement, et, d'autre part, que les perspectives de croissance de ces deux entreprises laissent présager de solides dividendes. Pour ADP, ensuite, le débat s'est beaucoup focalisé sur le fait de savoir s'il s'agissait de la privation d'un monopole ou bien d'infrastructures en situation concurrentielle. Si ce débat n'est pas tranché, tout au moins sommes-nous d'accord pour considérer qu'ADP est une infrastructure stratégique. Alors que, dans quelques jours, l'Europe va se doter d'un mécanisme de filtrage permettant d'évaluer le risque pour les infrastructures européennes stratégiques de tomber dans les mains d'actifs extra-européens, monsieur le ministre, il nous semble imprudent de laisser partir partir ADP sans en mesurer toutes les dimensions stratégiques. Or aucune garantie n'a été apportée sur les mécanismes de cessions des actifs à court, moyen et long termes qui peut dire, monsieur Yung, quel sera le sort d'un futur acquéreur privé, « opéable » une fois, deux fois, dix fois dans les 70 prochaines années ? Qui sera maître du jeu dans le ciel français ? Pour La Française des jeux, la FDJ, si le sujet de la santé et du rôle nécessaire de la régulation a été au coeur des discussions, c'est aussi le manque de réponse sur le financement de la filière équine et l'aménagement du territoire qui ont motivé notre avis. Pour autant, au sujet de ces deux sociétés, nos rapporteurs ont beaucoup travaillé pour améliorer, dans le cas d'ADP, le calcul des redevances aéroportuaires, ainsi que la régulation du secteur, et nous avons accepté la réforme de la fiscalité des jeux de la FDJ et des paris sportifs en ligne. Voilà quelques points, non exhaustifs, que le Sénat a améliorés au cours de ses travaux, ou sur lesquels il a marqué sa différence. C'est pour cette raison que le groupe Les Républicains votera le texte issu de nos travaux. Mais que dire du projet de loi dans sa globalité ? Il nous semble difficile aujourd'hui d'estimer correctement quel sera l'effet de ce texte protéiforme sur la croissance des entreprises. Si de nombreuses dispositions techniques sont attendues, il reste urgent, maintenant, de tenir les engagements sur la compétitivité. Les impôts de production ne baissent pas, la France reste championne d'Europe en matière de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques ; le déficit commercial se dégrade. Enfin, monsieur le ministre, les promesses de baisse de l'impôt sur les sociétés ne risquent-elles pas, à court terme, de se briser sur le mur jaune des réalités sociales.

ceux qui étaient pour le texte initial du Gouvernement ont voté contre, et ceux qui étaient contre le texte du Gouvernement ont voté pour. Au bout du compte, nous sommes dans une très grande confusion.

J'espère bien que certaines des propositions- je pense en particulier à tous les dispositifs d'encadrement et de renforcement des garanties autour des privatisations proposés par Jean-François Husson -pourront être reprises dans le texte définitif de la loi PACTE. Enfin, je veux rappeler quelques convictions et remettre quelques pendules à l'heure par rapport à ce que j'ai pu entendre. J'y insiste, ce texte est essentiel pour notre économie. d'abord essentiel pour les salariés. Je peux tout entendre, car nous sommes en démocratie, mais je ne laisserai pas dire que le projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises n'est pas une bonne nouvelle pour les salariés ! Ou alors, il faudra m'expliquer que la simplification de l'épargne salariale n'est pas une bonne nouvelle pour les salariés il faudra m'expliquer que le développement de l'actionnariat salarié n'est pas une excellente nouvelle pour les salariés il faudra m'expliquer que les garanties qui sont apportées aux femmes conjointes de collaborateurs, qui vont désormais bénéficier d'une protection renforcée, ne sont pas une bonne chose pour les salariés ; enfin, il faudra expliquer aux 10 millions de salariés qui vont enfin avoir accès à l'intéressement et à la participation grâce à la suppression

il va alléger un certain nombre de charges coûteuses ; il va nous remettre à niveau au regard des règles européennes pour tout ce qui est contrôle des comptes. En effet, je ne vois aucune raison pour que les entrepreneurs français aient des obligations en matière de certification des comptes plus strictes que celles de leurs voisins et concurrents espagnols, italiens, belges ou néerlandais. Nous remettons la compétitivité française à l'heure de l'Europe, en rappelant que les procédures françaises ne doivent pas être plus strictes que celles des concurrents européens. C'est une bonne chose pour les entrepreneurs également, puisque nous allons simplifier les seuils sociaux, en permettant à tous les entrepreneurs

d'abord, je rappelle qu'aucun dispositif n'est obligatoire pour les entrepreneurs dans ce texte. Tout est une faculté, rien n'est une obligation, parce que je pense que c'est ainsi que l'on fait progresser une société. Pour autant, croyez-moi, pour avoir discuté avec de jeunes entrepreneurs, avec de jeunes créateurs d'entreprise, que ce soit dans le domaine de l'artisanat, du commerce ou des start-ups techniques les plus pointues, je puis vous dire que tous veulent donner une raison d'être à leur société, parce que tous ont bien compris que l'entreprise ne se limite plus à la création de profit,

un sens à l'activité économique. Je me suis battu, avec Jean-Dominique Senard, avec Nicole Notat, avec un certain nombre de députés, avec des sénateurs, ici, pour que l'économie française prenne du sens : la raison d'être accordée aux entreprises, c'est du sens donné à notre modèle économique. Je pense, en dernier lieu, que ce texte est essentiel aussi pour l'innovation. C'est d'elle, monsieur Bourquin, que dépendra notre capacité à réindustrialiser notre pays. Je peux tout entendre, mais certainement pas que nous n'avons pas une politique industrielle pour notre pays, Agnès certainement pas que notre industrie continue son déclin, à un moment, monsieur Bourquin, où vous devriez partager avec moi la fierté des entrepreneurs industriels français, qui, pour la première fois depuis dix ans, recréent des emplois et rouvrent des entreprises dans nos territoires. nos territoires. À ces entrepreneurs, à ces industriels, qui se sont retroussé les manches, qui se sont battus, qui ont investi, digitalisé, robotisé, créé des emplois, même si ce n'est pas assez et s'il faut aller beaucoup plus loin, nous devons la reconnaissance d'avoir eu le courage de réindustrialiser nos territoires et notre nation. nation. Si nous voulons aller plus loin, il faut aussi donner à l'innovation davantage de perspectives. Tout ce qui figure dans le texte sur les liens entre recherche et entreprises est à cet

est une nécessité absolue pour financer le fonds pour l'innovation de rupture de dix milliards d'euros, qui nous permettra d'investir dans l'intelligence artificielle et dans les technologies nouvelles. Au XXI siècle, il y aura des vainqueurs et il y aura des vaincus ! Dans le camp des vainqueurs, vous aurez les nations qui auront investi pour l'innovation, celles qui auront la maîtrise de l'intelligence artificielle, des logiciels, des algorithmes, des données.

La séance est reprise. J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées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 mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui, en nouvelle lecture, le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et le projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions,

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, votre assemblée examine donc, en nouvelle lecture, les deux projets de loi qui constituent la réforme de la justice que je vous ai présentée au nom du Gouvernement au mois d'octobre dernier. Cette nouvelle lecture intervient après que le Sénat et l'Assemblée nationale n'ont pu trouver d'accord en commission mixte paritaire. Cet échec a traduit des divergences fortes entre les deux assemblées. Il faut constater qu'en première lecture votre commission des lois, puis votre assemblée avaient fait, pour l'essentiel, le choix de s'éloigner de la plupart des propositions formulées par le Gouvernement, propositions soutenues par la majorité de l'Assemblée nationale. Sans aller jusqu'à dire que deux projets s'opposaient, ce qui serait contraire à la réalité et sans doute trop caricatural, je constate que sur des questions essentielles, nous n'avons pas pu trouver de solutions communes. Je l'ai regretté au mois d'octobre, ici même, en observant que le Sénat avait fait le choix de ne pas partager les principales orientations contenues dans le projet initial du Gouvernement. Dès lors, les conditions d'un accord étaient presque impossibles à réunir. C'est la situation devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Pourtant, la volonté de donner à la justice les moyens d'accomplir son office est une ambition partagée par tous, je le sais. Sur chacune des travées dans cet hémicycle, comme au Palais-Bourbon, nous souhaitons que la justice dispose réellement des moyens de fonctionner de manière efficace sans rompre, en aucune manière, avec les principes qui la fondent.

J'entends bien que nous venons de loin- de très loin même !-, sur le plan budgétaire et que la justice doit disposer, c'est évident, à la fois de personnels plus nombreux et de moyens budgétaires plus importants. Je l'entends. Le Gouvernement l'a entendu lui aussi et y a répondu puisque ce budget progressera de 24 % sur cinq ans et permettra de recruter 6 500 emplois supplémentaires. la justice a également besoin d'être réformée. Il faut qu'elle s'adapte aux situations actuelles sans renier les principes fondamentaux qui la structurent. Réformer ne veut pas dire adopter une logique comptable ou une logique « d'économie de gestion », comme vos rapporteurs ont pu l'écrire. Ce n'est pas non plus déshumaniser la justice,

Ce qui me préoccupe, en réalité, c'est que les Français expriment une grande défiance à l'égard de la justice. Il est, pour moi, en tant que garde des sceaux, très difficile

Adapter notre justice, c'est avant tout lui permettre de répondre aux besoins des justiciables. Je mesure évidemment les attentes des professionnels avec lesquels j'ai beaucoup dialogué, à de nombreuses reprises.

nouveaux de compromis ont été apportés pour répondre aux demandes des avocats, des magistrats et des personnels de la justice.

Dans cette perspective, l'Assemblée nationale a d'ailleurs préservé un certain nombre d'avancées qui avaient été adoptées par le Sénat. Tel est le cas des garanties relatives aux services en ligne, qui ne pourront pas proposer des consultations juridiques sans le concours d'un avocat. Il en est de même pour le renforcement des obligations imposées aux plateformes. Je pourrais également citer la suppression de la représentation obligatoire devant les tribunaux paritaires des baux ruraux, l'inscription dans la loi des conditions d'expérimentation de la procédure de révision des pensions alimentaires, là où le Gouvernement demandait initialement une habilitation.

devant le juge d'instruction à la suite d'une plainte laissée sans réponse. Ce délai a été maintenu à trois mois en permettant au procureur de la République de solliciter du juge d'instruction un délai complémentaire de trois mois afin de poursuivre les investigations en cours. En matière d'alternative aux poursuites, l'actuelle limitation du champ d'application de la composition pénale aux délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans a également été maintenue. Des éléments destinés à mieux encadrer le rôle de la caisse d'allocations familiales ont été adoptés pour l'expérimentation, dont je parlais, que le projet de loi prévoit d'ouvrir en matière de révision des pensions alimentaires. Je pourrais citer, outre les dispositions qui ont clarifié certains points portant sur la répartition des contentieux spécialisés entre tribunaux judiciaires sur la base de projets locaux,

récapitulent des demandes souvent formulées par des professionnels du droit auxquelles il a été répondu, comme cela avait d'ailleurs été le cas sur plusieurs autres points lors de l'élaboration du projet de loi. Le texte a donc évolué très sensiblement. En revanche, le Gouvernement, et la majorité qui le soutient, a souhaité préserver les lignes de force de cette réforme. C'est ici que, pour l'essentiel, nous divergeons.

doute état. Je me contenterai de faire rapidement observer les éléments suivants. Sur la partie budgétaire, le Gouvernement a une approche à la fois ambitieuse et réaliste. Nous prenons en compte les contraintes d'ensemble de nos finances publiques et notre capacité concrète à réaliser un certain nombre d'équipements sur cinq ans, durée de la loi de programmation. Ce texte préserve d'ailleurs- je tiens ici à le souligner -les équilibres entre les moyens affectés aux juridictions judiciaires et ceux qui sont alloués à l'administration pénitentiaire. Sur la procédure civile, le projet que je défends a deux objectifs principaux : d'abord, simplifier l'accès du justiciable à la justice, ensuite, recentrer le juge sur son coeur de métier là où son rôle est essentiel, le juge doit être renforcé, notamment par les outils et les moyens qui lui sont alloués. J'avais d'ailleurs regretté, en octobre dernier, que votre assemblée soit revenue sur plusieurs mesures proposées par le Gouvernement. J'avais indiqué que je ne partageais pas un certain nombre de préventions du Sénat quant au recours au numérique et à la dématérialisation. Ces éléments me semblent constituer, au contraire, un très grand progrès en termes de modernité et de simplicité d'accès au droit et à la justice, si- et j'insiste sur cette condition -, les garanties nécessaires sont apportées pour que la justice demeure « humaine », au sens où elle nécessiterait elle nécessiterait la présence physique des magistrats et des personnels de justice. Le projet que je porte fournit ces garanties. Pour les assurer totalement, nous y avons d'ailleurs intégré un certain nombre de demandes exprimées par la profession d'avocat. Mais je défends aussi des positions réalistes, par exemple sur les plateformes qui constituent, je le crois, une évolution à la fois importante et inéluctable. Cela ne doit pas signifier que ces plateformes ne peuvent être en aucun cas régulées, mais il faut tenir compte de ce qu'est la réalité de l'économie du Net. C'est ainsi, me semble-t-il, que l'on apportera des garanties réelles aux justiciables qui auront recours à ces plateformes de plus en plus Sur la procédure pénale, nous avons aussi des divergences qui ont été exprimées à diverses reprises. Le texte que je propose ne constitue pas, contrairement à ce qui a pu être dit, une rupture avec les réformes qui se sont succédé depuis un quart de siècle. Ces réformes ont toujours entendu renforcer la capacité d'action des parquets pour adapter la réponse judiciaire à de nouvelles formes de délinquance mais en maintenant les droits de la défense et les garanties apportées aux justiciables. L'originalité de ma démarche ne vient donc pas de ce qu'elle inscrirait une rupture dans cette logique. Elle vient plutôt de ce que les propositions de simplification pénale contenues dans ce texte sont le fruit sont le fruit des propositions venues des acteurs de terrain, des policiers qui interviennent lors de la phase d'enquête, des magistrats du parquet et des magistrats qui ensuite jugent les litiges qui leur sont soumis. J'assume ma volonté de mieux protéger les Français tout en préservant la garantie des droits. Et ces garanties sont bien là, j'y ai veillé. Le Conseil d'État l'a amplement confirmé dans son avis. Au renforcement des pouvoirs des enquêteurs répond un contrôle des magistrats du parquet et du siège sur les actes d'enquête. Je rappelle que les magistrats du parquet sont avant tout des magistrats,

Le Sénat a très sensiblement modifié ce texte dans un sens qui m'a semblé, ainsi qu'à plusieurs observateurs, parfois éloigné des attentes exprimées par les juridictions, par les enquêteurs et par les justiciables. En tout état de cause, il faut que nous répondions à ce besoin clairement exprimé par nos concitoyens : le droit à la sécurité doit être pleinement garanti, dans des principes qui respectent l'État de droit. nous sommes, en outre, éloignés sur la partie consacrée aux peines. Les objectifs que nous poursuivons avec ce texte sont simples. Je le redis devant vous, l'idée, c'est que la peine de prison ne soit plus la seule peine peine de référence. Il faut que soient effectivement incarcérés ceux qui le méritent et pour lesquels c'est une nécessité, mais il faut punir autrement ceux pour qui la prison s'avérera inutile, désocialisante et source de récidives. C'est pourquoi j'ai proposé que les peines soient désormais réellement exécutées ; des peines également adaptées au profil de chaque délinquant, des lieux d'incarcération nouveaux et diversifiés, un suivi des détenus plus individualisé. Voilà ce que contient mon projet de loi

Vous ne souhaitiez pas, par exemple, faire du bracelet électronique une véritable peine autonome. De même, en créant une peine de probation autonome, le Sénat s'est inscrit dans les pas de la réforme ayant institué la contrainte pénale. L'évaluation de cette mesure montre qu'elle n'a malheureusement pas produit les effets attendus. Si je propose un sursis probatoire, mêlant la contrainte pénale et le sursis avec mise à l'épreuve, c'est précisément dans un souci d'efficacité et de souplesse, pour surmonter les difficultés rencontrées dans l'application de cette peine de contrainte pénale depuis sa création. Enfin, sur l'organisation des juridictions, mon objectif est, là encore, de simplifier la vie des justiciables en rendant plus lisible et plus compréhensible notre organisation, en maintenant tous les lieux de justice au nom du principe, absolument essentiel, de proximité pour la justice du premier degré. pour créer une juridiction unique de première instance, que vous aviez proposé d'appeler « tribunal de première instance » et que l'Assemblée nationale a dénommée « tribunal judiciaire ». En revanche, vous avez écarté la possibilité d'élaborer des projets locaux permettant de répartir quelques contentieux spécialisés entre les tribunaux judiciaires dans les départements comptant plusieurs tribunaux. Il en est de même pour une expérimentation identique qui concernerait deux régions comportant plusieurs cours d'appel.

a suscité des interrogations et des critiques. Je le comprends, mais je voudrais ici dire que le Gouvernement souhaite prendre ce dossier à bras-le-corps en s'appuyant sur le travail parlementaire qui a déjà été engagé sur ce sujet dans les deux assemblées. Le temps de la ratification sera pleinement employé pour que les deux chambres débattent de cette réforme et modifient le texte que le Gouvernement leur proposera, dans le sens qui leur semblera utile. Je suis absolument résolue à mener à bien cette réforme que deux majorités successives n'ont pas réussi à faire aboutir depuis plus de dix ans. sénateurs, que nous puissions trouver des terrains d'entente plus nombreux. Nous aussi ! Avant même la première lecture, j'avais fait part à M. le président de la commission des lois et à MM. les rapporteurs de ma volonté en ce sens. Les choix que vous avez alors exprimés et que vous avez réaffirmés depuis font que les conditions n'ont pas été réunies pour que cela soit possible. C'est ainsi. Le Gouvernement en prend acte et, comme les positions de chacun sont désormais claires, il ne déposera pas d'amendements pour revenir aux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale qui ont recueilli son accord. Cela nous éloigne, certes, pour un temps, mais je sais qu'à terme nous nous retrouverons pour que la justice puisse, en France, être mieux rendue au seul bénéfice des justiciables. La parole

Madame le président, madame le ministre, mes chers collègues, au nom d'Yves Détraigne et en mon nom ès qualités de rapporteur de la commission des lois, nous avons dix minutes pour vous rappeler rapidement

Je vous remercie, de ce point de vue, de bien vouloir respecter le travail de l'ensemble des collègues sur l'ensemble de ces travées, qui ont voulu appréhender

pouvons tout entendre, mais- je vous le dis très librement -nous ne pouvons pas tout accepter. Nous avons une vision différente de la vôtre,

afin que les personnes qui utiliseront ce dispositif soient protégées. Vous nous l'avez refusé ! Nous ne refusons pas toute

Nous avons proposé des évolutions en matière de droit commercial ; vous les avez refusées, alors que tout le monde était d'accord ! Nous avons également proposé un certain nombre d'évolutions en matière pénale.

Il n'est pas acceptable, pour la Haute Assemblée, de ne pas pouvoir lire et examiner ces textes. Je vous le dis très librement, très simplement, très directement, mais aussi, madame, très sincèrement.

Gardons ce qui peut être gardé ! Nous avons en revanche décidé de rejeter tout ce qui a été rajouté à l'Assemblée nationale : la réforme de l'ordonnance de 1945, la fusion des greffes des conseils de prud'hommes et des tribunaux d'instance, ou encore les modifications que vous avez faites sur les tutelles.

Nous avons enfin redit, très clairement, que les moyens budgétaires devraient être remis à niveau si l'on veut une ambition pour notre justice. Voilà ce qu'a fait la commission des lois, la semaine dernière et encore ce matin.

très haut niveau. Il y a un besoin d'organisation interne, de numérisation, bien évidemment, et de meilleure adaptation des procédures, mais cela se fera à l'unique condition que les justiciables y retrouvent leur compte et qu'ils puissent à tout moment rencontrer leur juge. Ainsi seulement, ceux qui doivent se défendre pourront le faire dans d'excellentes conditions. C'est le seul gage d'une justice acceptée, respectée, apaisante et garante du lien social absolument nécessaire dans notre pays qui est en train de souffrir de la douleur de la fraction. Bravo

Vous proposez un certain nombre de réformes, mais pour qu'une réforme puisse fonctionner, il faut un minimum de moyens ; or ces moyens ne sont pas présents. Il n'est pas possible

que les augmentations réalisées dans la décennie précédente et même au-delà. Rien n'est jamais assez pour la justice, j'en conviens avec vous, mais il faut aussi s'inscrire- je le répète -dans des contraintes globales.

Il faut faire évoluer nos de jugement et les secteurs sur lesquels nous intervenons, parce que cela répond aux attentes des justiciables et aux évolutions générales de notre monde. On ne peut pas se contenter d'abonder la justice en moyens sans jamais s'interroger sur la manière dont ces moyens sont utilisés. J'en viens à mon dernier point, que je ne développerai pas, parce que nous aurons l'occasion d'y revenir

Rien dans ce projet de loi, si ce n'est quelque fantasmagorie, ne vous permet de dire cela. Il faut un peu d'honnêteté intellectuelle quand on lit un texte. Je suis certaine que vous en avez, et c'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur cette motion.

Comme je l'ai dit en commission des lois, Mme Belloubet a réussi l'exploit de faire mieux que Mme Rachida Dati

comment ils sont utilisés et si l'on peut mieux les utiliser. Certes, mais regardez la place de la France en Europe ! Regardez les dépenses que nous consacrons à la justice

! Il faut faire un effort bien plus important que celui qui est prévu. D'ailleurs, quand vous aurez tenu compte de l'inflation sur la période de programmation considérée,

S'il y a bien un secteur qui est en péril alors qu'il est fondamental pour le fonctionnement de notre République, c'est bien celui-ci. Alors, madame la ministre, ne venez pas nous dire que votre projet est quelque chose de tout nouveau. Non ! C'est la suite de tout ce que l'on a connu jusqu'à présent, en pire

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le 30 janvier dernier, la commission des lois de notre assemblée eut l'heureuse initiative d'organiser une table ronde avec des représentants des syndicats, des associations et des conseils engagés dans l'action contre le projet de loi de réforme de la justice. Voyez-y la preuve, madame la ministre, de la rigueur intellectuelle du Sénat,

En tout domaine, le texte entérine un retrait et un affaiblissement de la justice dans le seul souci d'économiser des bouts de chandelles. » La justice de notre pays va mal les femmes et les hommes qui la portent au quotidien, quelles que soient leurs fonctions, sont à bout, usés par le flux tendu qui leur est imposé depuis des années. Des chiffres éloquents ont été rappelés le 30 janvier

faut pourtant rappeler que c'est l'administration pénitentiaire qui percevra, pour l'essentiel, les fruits de cette progression. Certes, il y a urgence, au vu de l'état déplorable des prisons françaises, mais n'est-il pas tout aussi urgent de permettre à la justice d'être plus efficace, non pas simplement pour condamner et pour sanctionner, mais aussi pour réinsérer et pour prévenir la récidive ? Désengorger les prisons requiert évidemment- pardonnez-moi cette lapalissade -que l'on cesse d'adopter des lois qui entraînent la surpopulation. Nous aurons l'occasion de constater une nouvelle fois, lors de l'examen des articles, que ce texte est truffé de mesures d'économie sur le rendu de la justice lui-même.

La dématérialisation à tout va, liée au développement de la procédure de conciliation, s'inscrit bien entendu elle aussi, sous un couvert grossier de simplification ou d'efficacité, dans cette logique d'austérité. La justice est ainsi traitée comme les autres services publics : on privatise, on externalise, on dématérialise, avec pour principales victimes non seulement les principes et les libertés, mais aussi, et surtout, les usagers et les personnels concernés. Sans reprendre mes propos de première lecture, je ne peux pas dissimuler un doute sur l'attitude de la majorité de la commission des lois dans ce débat. Bien entendu, comme nous l'avons souligné, l'intervention sénatoriale en matière civile est positive, en particulier dans le domaine de la conciliation et de la dématérialisation. Mais elle

Mais si ! Double peine, remise en cause du sursis, renforcement des conséquences de la récidive, et j'en passe ... le juge est préservé, mais poussé à toujours plus de répression, sans place aucune pour une réflexion alternative dont l'objectif serait moins de prison, plus de réinsertion, en un mot plus d'apaisement. Punir serait ainsi la seule fonction de la justice. Un tel dogme conduit tout droit à l'échec. En revanche, nous nous félicitons de la suppression par notre commission de l'article habilitant le Gouvernement à modifier l'ordonnance des mineurs de 1945 par voie d'ordonnance. Madame la garde des sceaux, nous espérons vivement que le Gouvernement se rangera à cet avis, renvoyant à un projet de loi cette nécessaire réflexion. Vous le savez, nous vivons un moment particulier de l'histoire de notre pays. Poussé par le mouvement des « gilets jaunes », le pouvoir organise un grand débat national. Peut-on concevoir que le service public de la justice, dont le bon fonctionnement garantit l'État de droit, ne soit pas l'un des sujets de cette discussion ? Tout à L'égalité face à la justice est un questionnement démocratique fort. Vous le savez tous et toutes ici, l'accès au droit n'est pas le même que l'on est riche ou pauvre. Les professions de la justice ne s'y sont pas trompées. Elles se sont lancées dans un mouvement d'ampleur, symbolisé par celui des robes noires, aux côtés des gilets jaunes ou des blouses blanches, pour défendre cet élément clé de la République qu'est la justice. La majorité sénatoriale a écouté ; c'est bien. Elle a en partie entendu. Mais, sur le fond, elle suit la voie du Gouvernement, en substituant de-ci de-là des possibilités à des obligations. nous estimons que ce projet ne laisse pas de place à la tergiversation ; il exige une opposition franche. Nous voterons donc

du projet de l'Assemblée nationale contre celui du Sénat, mais du projet du Gouvernement adopté par sa majorité à l'Assemblée nationale. Vous omettez de dire que toute l'opposition, de droite comme de gauche, s'est exprimée contre ce texte.

que le justiciable y ait de moins en moins recours. Or, précisément, dans une société démocratique, dans un État de droit, il est logique que chacun veuille faire valoir ses droits.

Mais ils ont insisté sur la nécessité d'une labellisation contrôlée. C'est ce que les rapporteurs ont proposé en première lecture sur la notion de certification. Pourquoi

La plupart des personnes entendues comme le résultat de nombre des consultations ont mis l'accent sur l'intérêt d'une peine de probation combinant ce qu'il y a de meilleur dans l'actuel sursis avec mise à l'épreuve qui est fréquemment prononcé et dans la contrainte pénale à laquelle, contrairement à ce qu'il était souhaité, il n'a pas été fréquemment recouru.

La République En Marche, le Président de la République, le Premier ministre et des ministres aller dans les grands débats citoyens pour, en fait, expliquer ce qu'ils font.

de la justice plutôt marqués à gauche déclarer que le Sénat avait mieux travaillé que l'Assemblée nationale ! Il est vrai qu'ils nous ont dit aussi que le Sénat les avait écoutés alors que l'Assemblée nationale ne semblait pas vouloir les entendre

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, je voudrais commencer par remercier nos deux rapporteurs et l'ensemble de nos collègues de leur investissement sur ce projet de loi très important. Avant même les mobilisations provoquées par l'examen du texte à l'Assemblée nationale, le Sénat avait identifié les sujets les plus problématiques et y avait apporté des réponses pour la plupart satisfaisantes et consensuelles. L'organisation L'organisation d'une nouvelle table ronde après l'échec de la commission mixte paritaire illustre la particulière implication de notre chambre sur le sujet. Nous n'ignorons pas que toutes les réformes sont difficiles à conduire, surtout quand elles affectent un grand nombre d'acteurs ayant des intérêts divergents. C'est le cas en matière de justice. Mais ici, ce sont tous les Français qui sont concernés. Notre devoir est de protéger les justiciables de manière équitable, de défendre les libertés individuelles et d'assurer la proximité du service public de la justice. Les préoccupations peuvent d'ailleurs sensiblement varier selon que l'on se situe en zone urbaine ou en zone rurale. Avec la complexification des parcours de vie familiaux, professionnels et géographiques, notre réflexion doit se poursuivre. On ne peut pas se cantonner dans une attitude seulement conservatrice consistant à vouloir maintenir l'existant. Ce n'est pas la position de notre Haute Assemblée. Dès 2017, l'investissement de l'ensemble de l'hémicycle sur la proposition du président Bas a montré notre volonté de prendre à bras-le-corps tous les défis qui s'imposent aux justiciables et aux professionnels du droit, malgré plusieurs points de désaccord. L'article 1 du projet de programmation budgétaire est certainement le plus important. La justice souffre d'un manque d'investissement substantiel. L'effort budgétaire consenti, qu'il soit de 20 % ou 30 % sur quatre ans, devrait permettre d'améliorer les conditions de travail dans les juridictions. Quand on voit les résistances que le reste des dispositions suscitent, on n'est pas loin de se demander s'il n'aurait pas fallu se limiter à cet engagement budgétaire à droit constant ou presque, avant d'ouvrir les chantiers de la justice. À l'avenir, il serait peut-être sage de s'imposer comme doctrine de n'ouvrir que des chantiers que l'on est certain de pouvoir sereinement conduire à leur terme. En effet, aucun aspect de la justice n'échappe à ces projets de loi développement de la médiation et de la conciliation, justice civile, affaires familiales, plateformes de services juridiques en ligne, justice administrative, procédure pénale, droit pénal et même justice pénale des mineurs, que vous proposez de réformer par ordonnance. Par la multitude des sujets qu'ils abordent, les effets escomptés de ces textes sont devenus impossibles à anticiper. Nous regrettons particulièrement que la réforme pénale n'ait pas fait l'objet d'un texte distinct, en lien avec les très nombreuses réformes de sécurité intérieure qui se sont succédé après les attentats de 2015. Car, dans ce domaine, la défiance s'ajoute aux manques de moyens. Là plus qu'ailleurs, il est dangereux de vouloir réformer sans s'assurer que des garanties élémentaires seront effectivement observées. Je pense en particulier au développement des techniques spéciales d'enquête, qui font reposer la protection des libertés individuelles sur un contrôle aujourd'hui purement formel des juges. Parmi les points de consensus dans notre chambre- le sujet inquiète également de nombreux collègues députés -, il y a évidemment la question de la carte judiciaire et l'inscription de la justice dans l'espace national. Nous avons pris acte de votre engagement personnel et sincère à maintenir des lieux de justice à bonne distance de tous les justiciables, madame la garde des sceaux. Mais notre rôle est de nous assurer que cet engagement vous survivra sur du plus long terme. À ce titre, la rédaction adoptée par la commission des lois offre de meilleures garanties que le texte résultant des travaux de l'Assemblée nationale. Sur la question de la dématérialisation, de la même manière qu'il faut veiller à se départir de tout conservatisme, je crois qu'il est nécessaire de relativiser les retombées potentielles d'une transformation numérique des relations entre la justice et le justiciable. Il faut bien le reconnaître, il existe aujourd'hui un fantasme administratif transversal selon lequel le recours aux nouvelles technologies serait la solution à tous les problèmes. Ce projet de loi n'y échappe pas. S'agit-il de rendre justice ou, pour l'administration, de limiter ses rapports avec les justiciables ? S'agit-il d'instituer une nouvelle intermédiation fragilisant l'accès au juge ? Le dernier rapport du Défenseur des droits dénonçant les liens entre la dématérialisation et les inégalités d'accès aux services publics abonde dans notre sens. De la même manière, il est probable que les plateformes numériques en ligne serviront de miroir aux alouettes pour les justiciables les moins bien informés. Les autres continueront de solliciter des juges. Sur d'autres questions, comme la lutte contre les violences sexuelles et la création d'un tribunal criminel départemental, nous avancerons également sans dogmatisme. C'est dans cet esprit que nous abordons cette nouvelle lecture. La parole

Partout, dans la fonction publique, on pousse et on incite à la mobilité des fonctionnaires, parce que c'est un gage d'expérience, de diversification et de meilleure administration. Dans l'administration de la justice, la mobilité répond également à cette finalité. Mais, pour la justice, je crois qu'il y a une autre nécessité dans la mobilité pour la justice, je crois qu'il y a une autre nécessité dans la mobilité : celle de l'indépendance des juges par rapport au contexte local.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes de nouveau réunis pour l'examen de ce texte d'une importance capitale. La justice est, certes, un service public, mais c'est surtout l'incarnation d'un pilier de la démocratie, du « troisième pouvoir » décrit par Montesquieu. Faute d'effectifs suffisants ou de respect vigilant de certains principes, elle peut faire basculer un régime démocratique, et également broyer des vies. Il importe donc de se montrer particulièrement vigilant lorsqu'il s'agit d'en modifier les règles ou le fonctionnement. C'est un pouvoir régalien qui doit être accessible à tous. Son efficacité et son organisation ne peuvent pas se mesurer à l'aune d'un prisme purement comptable. En première lecture, le Sénat a apporté des évolutions avisées et nécessaires à ce projet de loi. On peut évoquer ici une trajectoire budgétaire ambitieuse, avec une création de 13 700 emplois là où- il faut bien le dire -le Gouvernement n'en prévoit que 6 500. Le budget proposé par le Gouvernement est, certes, important, mais son affectation concernant les juridictions est loin d'être satisfaisante. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été rappelés par mes collègues. Dans Dans l'objectif de garantir l'équilibre de la procédure pénale et de limiter le renforcement excessif des pouvoirs du parquet, le Sénat a veillé à ne pas marginaliser le juge d'instruction et à maintenir la collégialité des travaux de la chambre de l'instruction. La collégialité est une garantie en matière d'échanges, d'ajustements, d'examen concerté et minutieux des cas d'espèce, en bref d'impartialité et de considération de la situation du justiciable. Nous savons tous combien, particulièrement dans le domaine pénal, une affaire apparemment simple peut se révéler complexe. Nous savons aussi que les juges sont surchargés. À l'évidence, comme pour tout un chacun, leur attention ne peut pas être aussi aiguë à la vingtième ou trentième affaire de la journée qu'à la première. J'aurais pour ma part souhaité une réduction des formations à juge unique. L'inflation des missions dévolues au parquet est une caractéristique majeure du texte. Sur le plan de l'efficacité et de la rapidité- c'est à l'évidence le premier objectif du projet de loi -, une telle orientation laisse dubitatif.

Un fait est certain : la logique inquisitoire se substitue insidieusement à la logique accusatoire, et les droits de la défense se font de plus en plus timides. Accroître les pouvoirs du parquet, c'est aussi occulter le fait que, quelles que soient les compétences et l'évidente valeur professionnelle de ses membres, celui-ci ne constitue pas une « autorité judiciaire » au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La France a déjà été condamnée plusieurs fois. La situation ne pourra pas s'améliorer tant que des garanties supplémentaires d'indépendance statutaire n'auront pas été apportées par une révision constitutionnelle. Tant qu'une telle révision n'aura pas été adoptée, il ne sera pas raisonnable de continuer à confier au parquet des pouvoirs toujours plus importants et de le rendre seul décisionnaire de l'utilisation de techniques d'enquête les plus intrusives qui soient pour la vie privée et les libertés individuelles. techniques, jusqu'alors réservées au terrorisme et à la criminalité organisée, seront exerçables à l'encontre de tout justiciable soupçonné d'un délit quel qu'il soit, même le plus mineur. La question des moyens et de leur affectation est essentielle pour offrir à nos concitoyens une justice de qualité, une justice accessible offrant protection et garanties d'impartialité. Elle ne saurait en aucun cas trouver une solution dans de simples réorganisations : suppression de tribunaux d'instance, déjudiciarisation ou encore dématérialisation débridée des procédures. Les crédits dévolus au programme « Justice judiciaire » seront-ils suffisants pour redresser le service public de la justice ? Non, sauf à réduire drastiquement son rôle auprès des citoyens. C'est malheureusement le chemin qui semble être pris : déjudiciarisations coûteuses pour le contribuable ; règlements amiables de litiges en ligne non sécurisés, ce qui laissera les plus vulnérables de nos concitoyens être la proie des pires escrocs ; plaintes en ligne, alors que, pour information, presque le quart des Français ne sait pas utiliser l'outil numérique- je crois que le chiffre exact est 23 disparition progressive des audiences de conciliation ; disparition programmée des jurés, et ne parlons même plus du juge de paix, passé, lui, aux oubliettes. L'individu, le justiciable, existe-t-il encore face à cette- oui, madame la garde La question se pose. S'agit-il d'une justice à deux vitesses ou d'une justice en perte de vitesse ? À l'évidence, des deux. Les professionnels du droit sont très inquiets. Le 29 janvier dernier, la commission des lois du Sénat a invité à débattre les représentants du monde judiciaire : avocats, bâtonniers, magistrats et fonctionnaires des greffes. La Confédération nationale des avocats, par l'intermédiaire de son président, M. Spitz, a souligné l'unanimité des professionnels du droit pour défendre l'intérêt du justiciable. Cette unanimité est en effet rare, très inhabituelle. M Marie Aimé Peyron, bâtonnier du barreau de Paris, a salué le travail sénatorial sur le rééquilibrage entre les droits des victimes et les droits de la défense en matière pénale, et lourdement insisté sur le cruel manque de moyens humains et financiers. L'affectation des moyens laisse le monde des juridictions bien à l'écart de la manne budgétaire, les moins bien lotis étant les greffiers, grands oubliés de la réforme, ainsi que le personnel affecté au réseau judiciaire de proximité. Il n'y a pas de hasard. Jérôme Gavaudan, président de la Conférence des bâtonniers, et Katia Dubreuil, présidente du Syndicat de la magistrature, ont dénoncé la fusion des tribunaux comme la fin des juridictions de proximité.

Face à ce projet de loi, contesté et profondément rejeté par l'ensemble des professionnels du droit, je salue la démarche du président de notre commission des lois, M. Philippe Bas : tenter jusqu'au bout d'obtenir un compromis avec vous, madame la garde des sceaux. Je salue également encore une fois les professionnels du droit, qui ont su faire fi d'intérêts parfois très divergents pour s'unir dans la défense de la justice et du justiciable. La réforme de la justice, ses enjeux et les obstacles que rencontrent chaque jour les justiciables et les professionnels doivent faire partie intégrante du grand débat national. Pourtant, cette réforme essentielle tant sur le plan pratique que sur le plan fondamental de nos principes démocratiques en est exclue ! Exclue parce que la procédure législative est en cours et qu'il ne faut toucher à rien de ce qui est engagé. C'est inouï, c'est ubuesque : c'est tout simplement antidémocratique Tout est encore possible, vous pouvez encore entendre le Sénat, madame la garde des sceaux, vous pouvez encore entendre les professionnels du droit et surtout entendre les citoyens. Ce sont eux les premiers concernés et ils doivent pouvoir, à l'heure de ce grand débat national, donner leur avis L'Assemblée nationale a d'office quasiment rétabli le texte initial du Gouvernement, en balayant comme billevesées les modifications apportées par le Sénat. Il est ici nécessaire d'insister sur les difficultés croissantes des deux chambres à s'entendre sur un texte commun ou plutôt sur le refus du groupe majoritaire de l'Assemblée nationale à accepter un point de vue différent de celui du Gouvernement. Le nombre de commissions mixtes paritaires conclusives est en diminution drastique depuis juillet 2017. Depuis 1958, la règle a toujours été l'accord entre nos deux assemblées. Entre 1958 et octobre 2017, seulement 12 % des textes ont été adoptés par la procédure dite du « dernier mot » à l'Assemblée nationale.

Les commissions mixtes paritaires ont pour objet de permettre l'avènement du jeu démocratique. Le bicamérisme est essentiel parce qu'il reflète l'accord entre l'avis d'une chambre dédiée au pouvoir exécutif et celui d'une chambre qui ne dépend pas de lui, entre la France du moment d'une élection présidentielle et celle d'une élection à mi-mandat. Enfin, le bicamérisme est issu de l'essence même de la démocratie et de la théorie des contre-pouvoirs. Les corps intermédiaires, les contre-pouvoirs sont essentiels à la République, ne pas les entendre est extrêmement dangereux. Entendez les voix qui s'élèvent, madame la garde des sceaux, cette unanimité doit vous alerter. Aujourd'hui, nous sommes responsables pour demain.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui, en nouvelle lecture, le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et le projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions, les commissions mixtes paritaires du 13 décembre dernier n'ayant pas été conclusives. Au vu du texte résultant des travaux de l'Assemblée nationale et compte tenu de la forte hostilité exprimée au sein des milieux judiciaires contre la réforme telle qu'elle est envisagée par le Gouvernement, la commission des lois a organisé à la fin du mois de janvier une table ronde avec les représentants des avocats, des magistrats et des fonctionnaires de greffe. Trouver des solutions d'avenir, nourrir le dialogue, tels étaient les objectifs de cette initiative visant à écouter les inquiétudes exprimées par les professionnels de la justice. Je me félicite donc de cette volonté de travailler à la recherche de convergences, mais également de se situer au-delà des clivages. C'est cet esprit de compromis et de dialogue qui permet au Sénat d'avoir des travaux de grande qualité ! C'est précisément cet esprit qui a conduit la commission à conserver les modifications et ajouts de l'Assemblée nationale lorsque ceux-ci s'avéraient pertinents et ne soulevaient pas de difficulté de principe. C'est toujours cet esprit qui a permis de prendre en compte les craintes du monde judiciaire et des territoires. La commission a bien entendu les interrogations relatives à la pérennité de la carte judiciaire. En tant que rapporteur pour avis sur les crédits du programme « Administration pénitentiaire », je me réjouis particulièrement que la commission ait rétabli la trajectoire budgétaire de la mission « Justice », telle qu'adoptée par le Sénat en première lecture. Elle prévoit une augmentation des crédits de 33,8 % entre 2017 et 2022, et la création de 13 700 emplois. La programmation du Gouvernement, rétablie par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoyait une progression des crédits de 23,5 % et la création de 6 500 emplois sur la même période. Or cela paraît bien insuffisant pour assurer le redressement budgétaire des juridictions et de l'administration pénitentiaire. En effet, cette trajectoire doit également permettre de mettre en oeuvre le programme de construction de 15 000 places supplémentaires de prison, figurant dans les engagements de campagne du Président de la République. En matière de justice civile, la commission a largement rétabli le texte adopté par le Sénat en première lecture, avec l'intention d'améliorer les procédures et de mieux protéger les personnes les plus fragiles. Elle a en effet conforté et mieux encadré le recours aux modes alternatifs de règlement des différends, dans l'intérêt des justiciables. Elle a notamment rétabli l'exigence de certification obligatoire par le ministère de la justice des services en ligne de résolution amiable des litiges et d'aide à la saisine des juridictions, dans l'objectif d'imposer des garanties pour les justiciables pouvant recourir à ces services. Elle a ensuite choisi de maintenir la phase de conciliation judiciaire dans la procédure de divorce contentieux, compte tenu de son intérêt pour les parties. Elle a également veillé à mieux protéger les personnes les plus vulnérables en préservant le rôle protecteur du juge. Enfin, s'agissant de la réforme de l'organisation judiciaire, si le regroupement du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance cristallise à lui seul une large part de l'opposition du monde judiciaire, qui craint un éloignement pour le justiciable et la suppression de sites judiciaires, la commission a repris les garanties que le Sénat avait déjà apportées en première lecture, et qui sont susceptibles d'apaiser certaines des craintes exprimées. Parmi ces garanties, je citerai la suppression de la possibilité de spécialiser certains tribunaux en matière civile et pénale lorsqu'il existe plusieurs tribunaux au sein d'un même département. Je fais également référence à la fixation au niveau national d'un socle minimal de compétences des chambres détachées remplaçant les tribunaux d'instance situés en dehors du siège du nouveau tribunal unifié, afin d'éviter qu'elles ne soient définies au cas par cas, de façon trop trop limitée ou résiduelle, des compétences supplémentaires pouvant en outre leur être attribuées par les chefs de cour sur proposition des chefs de juridiction. Je veux aussi mentionner la création d'un dispositif d'encadrement de toute modification de la carte judiciaire, laquelle relève de la compétence du pouvoir réglementaire, comportant une évaluation, au vu des observations présentées par les chefs de cour ainsi que par le conseil départemental, dont il serait rendu compte dans un rapport public, et sur la base de critères objectifs préexistants. Concernant le régime des peines, je me réjouis particulièrement que la commission ait rétabli le texte que le Sénat avait voté en première lecture, lequel prévoyait notamment une importante refonte du système de l'aménagement des peines, de façon que la peine prononcée soit en principe la peine exécutée Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ces deux textes ainsi modifiés par la commission des lois. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous avons tenté de nous accorder avec l'Assemblée nationale sur des textes communs de réforme pour la justice le 13 décembre dernier. Malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus et les commissions mixtes paritaires ont échoué ... Hélas ! ... malgré le formidable travail des rapporteurs, ... En effet. ... notamment. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui pour les examiner en nouvelle lecture. Alors même que ces deux textes ont fait l'objet de larges consultations, qu'ils ont évolué au cours des discussions entre la Chancellerie et le milieu judiciaire, un mouvement de contestation semble s'être cristallisé. La commission des lois a, pour chercher à sortir de cette impasse, organisé le 30 janvier dernier une table ronde avec les représentants des milieux judiciaires, qui a été suivie par votre audition, madame la garde des sceaux. Si je n'ai pu physiquement y assister, j'ai suivi ces discussions avec grand intérêt grâce à la captation vidéo qui a été retransmise sur le site internet du Sénat. Je voudrais néanmoins effectuer une correction, qui a son importance, quant aux termes choisis par notre commission. Il ne s'agissait pas, comme j'ai pu le lire, de « tenter de renouer le dialogue », car celui-ci n'a jamais cessé. Vous avez entrepris, madame la garde des sceaux, un grand tour des juridictions françaises afin de présenter votre réforme et vous avez, depuis le printemps, régulièrement rencontré les avocats. Vous vous êtes d'ailleurs rendue à la rentrée du barreau de Paris et, très récemment, à l'assemblée générale statutaire de la Conférence des bâtonniers. Si ces échanges n'ont pas répondu à l'ensemble des attentes des acteurs de la justice, il est inexact de dire que votre position n'a jamais pu être infléchie et que vous vous êtes montrée hermétique aux arguments qui vous ont été opposés. Au contraire, ces échanges nourris ont permis de faire évoluer sensiblement les textes examinés par notre assemblée. Je pense, notamment, au renforcement des obligations des plateformes numériques ; à la simplification de la procédure de divorce contentieux qui permet de ne pas causer le divorce dès l'introduction de la procédure à la généralisation des règles protectrices en matière de perquisitions effectuées dans le cabinet d'un avocat, à son domicile, dans les locaux de l'ordre des avocats ou des ou encore à l'encadrement du rôle des CAF dans la révision des pensions alimentaires en rendant possible la suspension provisoire de la décision et le recours devant un juge. Je pense également à la réforme des ordonnances d'injonction de payer, qui vise à centraliser le traitement des injonctions de payer aux fins d'une meilleure efficacité. Paradoxalement, ces compromis ont parfois été qualifiés de reculs du Gouvernement. C'est à n'y rien comprendre ! Concernant l'organisation judiciaire, vous n'avez jamais cessé de tenter de rassurer les professionnels qui redoutent légitimement que la réorganisation des juridictions ne se traduise par la fermeture de sites, en martelant que vous maintiendrez les hommes, les lieux et les compétences existants. Lorsqu'il existe plusieurs TGI, le texte offre, je dis bien « offre », la possibilité aux juridictions de spécialiser les contentieux techniques et- et non pas ou, car la conjonction de coordination a ici son importance -de faibles volumes, ce qui exclut les contentieux de masse. Face à la crainte légitime d'une « robotisation », d'une « déshumanisation » de la justice que pourrait induire la dématérialisation des procédures, vous avez précisé que le numérique ne viendra pas se substituer, mais viendra s'ajouter à l'accueil physique. Ainsi, pour les justiciables peu familiarisés avec les nouvelles technologies ou habitant dans une zone qui les prive d'un accès internet de qualité, un guichet d'accueil physique sera maintenu dans chaque lieu de justice. La numérisation présente un intérêt tant tant pour les victimes, qui peuvent être intimidées par un dépôt de plainte dans un commissariat, que pour les praticiens du droit, lesquels se heurtent souvent- croyez-en mon expérience -à des temps d'attente téléphonique particulièrement longs pour obtenir parfois la seule confirmation qu'un acte a bien été enregistré. L'Assemblée nationale a procédé à des améliorations intéressantes telles que l'extension des possibilités d'anonymisation des policiers et gendarmes dans les procédures ou encore le dossier entièrement numérique dans le cadre de la procédure pénale. En revanche, si comme nombre de mes collègues, je suis favorable à réformer la justice des mineurs afin de la rendre plus lisible pour les professionnels et les justiciables, et de renouer avec son esprit fondateur, tendant à faire primer l'éducation sur la répression, je regrette néanmoins que vous ayez choisi de passer par la voie de l'ordonnance pour ce faire. J'aurais préféré que le Parlement ne soit pas ainsi dessaisi. Je forme Je forme malgré tout le voeu que la réforme que vous envisagez tiendra compte des travaux de nos assemblées sur ce sujet- je pense, notamment, au rapport de la mission d'information sur la réinsertion des mineurs enfermés ou à la mission en cours à l'Assemblée nationale sur la justice des mineurs et qu'elle sera menée en toute transparence, avec le concours des parlementaires. Je vous fais d'ores et déjà savoir que nous voulons y être associés. Pour conclure, malgré nos divergences d'opinions, j'avais formulé, en première lecture, le voeu que le débat se poursuive à l'Assemblée nationale, parce que nous souscrivons tous à cet objectif d'une justice plus simple, plus rapide et plus efficace. Dans ce même esprit, j'espère encore que des compromis raisonnables puissent être trouvés avec nos collègues de l'Assemblée nationale sur certains sujets comme le dispositif de certification obligatoire des plateformes de résolution amiable des litiges, la suppression de l'extension de l'obligation de tentative de règlement amiable préalable préalable à toute saisine du juge en matière civile ou la limitation de l'extension des techniques spéciales d'enquête. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe La République En Marche s'abstiendra sur ces textes. La parole est à Mme Sylviane Noël. Madame la

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, ce projet de loi entend répondre au besoin d'équité de notre société, qui dénonce avec pugnacité la lenteur de la justice, et parfois la distance qu'elle observe par rapport aux réalités vécues par nos concitoyens. Pourtant, force est de constater que cette réforme ne tient absolument pas compte des caractéristiques de certaines zones géographiques. Car si la France est une et indivisible, elle n'est pas uniforme ! Oui, la France est un grand pays fort de la diversité de ses territoires où tout ne fonctionne pas comme à Paris Dans le contexte de crise que nous traversons, le Gouvernement assure avoir saisi la portée de la colère des Français. Ces mêmes Français qui se retrouvent dans l'incompréhension face à toutes les réformes qui ne vont résolument pas dans leur sens. Prenons la modification de la carte judiciaire. Elle est vécue comme un coup de grâce porté au rôle pourtant prépondérant que joue l'institution judiciaire dans nos territoires. Par ce texte, notamment au travers de l'article 53, les juridictions se retrouveront demain vidées d'une grande partie de leurs compétences puisque vous entendez fusionner les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance pour créer un seul tribunal de première instance dans chaque département. Vous centralisez l'activité judicaire alors qu'il conviendrait dans certaines zones de maintenir une proximité qui permettrait de conserver un lien cher avec nos administrés. Cela n'est pas sans conséquence. Par exemple la Haute-Savoie compte actuellement trois tribunaux de grande instance : Bonneville, Thonon et Annecy. Ils devront, si cette loi est adoptée, transférer leurs compétences au tribunal de première instance, qui traitera les matières dans des pôles dédiés, et deviendront par ailleurs des centres d'accueil qui permettront aux justiciables d'entamer toutes les étapes préalables à l'audience. Or c'est oublier que dans ces départements de montagne, les distances ne se comptent pas en kilomètres, mais en temps de parcours. Ce sont des territoires reculés, enneigés une grande partie de l'année, où il faut parfois faire plusieurs heures de voiture pour atteindre une destination éloignée de quelques kilomètres ! Ce sont des départements qui, malgré leur éloignement, sont pourtant des territoires extrêmement vivants et qui connaissent une activité judiciaire intense. Comme en Haute-Savoie, territoire pour le moins atypique, dont l'activité judiciaire n'est pas en reste puisque ce département enregistre à la fois la plus forte croissance démographique de notre pays, la plus forte concentration mondiale d'entreprises de la mécatronique, compte plus de lits touristiques que d'habitants permanents et est de surcroît doublement frontalier avec la Suisse et l'Italie. Pour ces territoires, un tel schéma de délocalisation de certains contentieux entraverait considérablement l'accès des citoyens à la justice puisque ces derniers devront parcourir plus de 100 kilomètres pour se rendre à une audience. Au-delà de l'aspect géographique, la réalité est bien entendu fonctionnelle. Les professionnels de la justice, les élus locaux, dont je suis l'un des porte-parole dans cet hémicycle, s'inquiètent, eux aussi, de pouvoir garantir une certaine proximité de leurs actions, d'autant que l'efficacité et la performance de ces juridictions sont unanimement reconnues. Comment sauront-ils rester à l'écoute des justiciables, d'une part, en les accueillant physiquement au sein des services d'accueil unique du justiciable et, d'autre part, avec des moyens qui seront demain dématérialisés ? Comment assureront-ils un contact décent au cours des diverses procédures, de l'audience jusqu'à la décision finale, afin de faciliter les démarches de nos administrés ? Comprenez, madame la ministre, que dans la période difficile que nous traversons, la justice ne saurait être un facteur supplémentaire de fracture sociale et territoriale. À l'instar de Joseph Joubert qui aimait à rappeler que la justice est le droit du plus faible, souvenons-nous que la justice doit être plus que jamais un point de cohésion et d'équité nationale ! La parole

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je veux d'abord dire toute ma reconnaissance à nos rapporteurs qui, avec beaucoup de persévérance, ont poursuivi la tâche pour donner jusqu'au bout toute leur chance aux mesures d'apaisement et de raison proposées par le Sénat. Au moment de prendre la parole, je veux exprimer le sentiment d'un certain gâchis. Après l'échec de la commission mixte paritaire, nous avons renoncé, ce que nous avons confirmé par notre vote aujourd'hui,à adopter une motion tendant

du plus large accord possible sur les axes fondamentaux de la réforme avec les professions de justice. Vous me rétorquerez que nous nous sommes élevés un peu au-dessus de notre condition de sénateur en prétendant apporter notre secours au Gouvernement, qui se heurte aujourd'hui de bons Samaritains ! ... puisque la table ronde que nous avons organisée il y a quinze jours a fait apparaître une très large convergence des avocats, des syndicats de magistrats et des syndicats de personnels des greffes autour d'un certain nombre de demandes. Madame la garde des sceaux, les professions de justice ont des attentes. Chacun est conscient de la nécessité de réformer. Nous partageons le même diagnostic sur la situation

de trouver des solutions consensuelles ne soit pas saisie. Cette impasse n'est pas une impasse législative. Bien sûr, vous disposez, madame la garde des sceaux, d'une majorité à l'Assemblée nationale pour voter votre texte, car les institutions de notre pays apportent au Gouvernement la stabilité dont il a besoin : un Président de la République tout-puissant, un gouvernement qui lui est naturellement subordonné et une Assemblée dans sa majorité, qui a été désignée peu après l'élection présidentielle pour soutenir le Président de la République. C'est donc seulement ici, au Sénat, que vous pouvez trouver les voies d'un dialogue avec d'autres que ceux qui vous soutiennent, mais qui sont de bonne volonté pour permettre à la justice d'échapper au clivage partisan, ce qui est notre souhait le plus profond. Nous avons vu récemment quels sont les résultats d'une méthode de gouvernement pouvant se résumer par la volonté d'un passage en force quand on est sûr d'avoir raison. raison. Mais si le Gouvernement a une pédagogie, il lui manque une capacité de dialogue. Nous étions nombreux à penser que les leçons de l'expérience récente allaient servir et que la justice pourrait être le terrain d'expérimentation d'une autre méthode de gouvernement.

vous rappeler que la période durant laquelle les alternatives à la prison- c'est-à-dire le bracelet électronique -se sont le plus développées, c'est la fin du mandat du Président Sarkozy ? Depuis, calme plat ! Cependant, il ne il ne suffit pas de développer les alternatives à la prison pour s'accommoder de la situation de surpopulation carcérale que nous connaissons. Si les magistrats prononcent aujourd'hui des peines de prison, ce n'est pas simplement parce qu'ils préfèrent la prison c'est aussi parce c'est aussi parce que les alternatives à la prison ne bénéficient pas des moyens nécessaires à leur développement. Nous en arrivons alors à notre deuxième point de divergence, qui est celui du budget. Certes, dans cette

après le prochain quinquennat. Il s'agit à nos yeux d'un point important. Au fond, une vraie loi de programmation doit commencer dans les trois mois qui suivent l'élection présidentielle, sinon cela n'a guère de sens ! Vous n'avez plus aujourd'hui que deux lois

des moyens de la justice, en ancrant cette évaluation dans une comparaison européenne. Or nous sommes vraiment très en retard et il convient de mettre les bouchées doubles

Enfin, nous ne sommes pas d'accord avec le parquet national antiterroriste et nous regrettons que ce texte ne contienne pas de disposition pour assurer la pérennité du financement de l'aide juridictionnelle, qui est la condition

Vous avez purement et simplement voulu rétablir votre texte initial et faire l'économie du dialogue avec le Sénat. De la même façon, vous selon moi de manière excessive, l'économie d'un dialogue approfondi avec les professions de justice au moment où elles vous demandent d'infléchir votre réforme.

vous auriez pu faire un effort sur la certification des plateformes proposant des possibilités de conciliation sur internet. Ce n'eût pas été de votre part un effort disproportionné

sur le refus d'informer l'avocat sur des perquisitions, sur la comparution différée, sur l'accès au dossier par l'avocat, vous avez pris des mesures qui vont toutes dans le même sens, et qui n'est pas celui des garanties offertes à nos concitoyens face au ministère public. Quant à l'organisation judiciaire, c'est évidemment pour nous un sujet de vive préoccupation. Au fond, nous vous demandions de sécuriser les chambres détachées en prévoyant la création d'un juge chargé des contentieux de proximité, une garantie de localisation des emplois pour les fonctionnaires de greffe dans ces chambres détachées et la définition d'un socle minimal de compétences au niveau national pour ces chambres. De la sorte, vous auriez pu tenir en échec tous ceux qui affirment- peut-être à tort -que vous préparez la suppression de lieux de justice, alors que vous proclamez régulièrement qu'il n'en est rien et que vous voulez conserver ces lieux de justice. Donnez-nous des gages de cette volonté de les conserver et nous pourrons vous soutenir.

Monsieur le président, je suis obligée de vous demander de conclure. Alors, je conclus. Aujourd'hui, un simple décret peut modifier la carte des tribunaux.

Que demandent les associations de victimes que j'auditionne ? Elles demandent les mesures que nous avons prises dans le texte. Je pourrais ainsi continuer longtemps ... Il y a dans ce texte des éléments-

à travers lui une réforme absolue et générale de la justice. Ce texte a une ambition claire : faire évoluer la justice de notre pays. Il ne prétend pas, à lui seul, embrasser toutes les toutes les évolutions qui seraient envisageables pour la justice en France. Il faudra, bien sûr, monsieur le sénateur Masson, que nous soyons attentifs à la gestion des ressources humaines. Vous évoquiez la question de la mobilité des magistrats. C'est une vraie question, même si je ne l'entends pas exactement dans le sens que vous avez évoqué.

Je regrette que nous n'ayons pas pu parvenir à un accord, mais je suis persuadée que, lors de l'application effective du texte, nous saurons retrouver des capacités de dialogue.

sur la justice. On ne peut pas, d'un côté, organiser un grand débat sur tout le territoire pour tenter de recréer du lien avec les citoyens et, dans le même temps, entamer une réforme de la justice, décriée par de très nombreux professionnels qui manifestent et alertent

» Que fait cette réforme de la justice ? Elle éloigne la justice d'un citoyen qui souffre de cette déshumanisation progressive de la société. Elle porte atteinte à l'oralité des débats dans la mesure où le tribunal criminel départemental prendra en charge une partie des affaires actuellement traitées par les cours d'assises et ne sera pas composé d'un jury populaire tiré au sort. C'est dommage, à l'heure même où le peuple demande à participer davantage à la vie de la cité. De plus, la spécialisation des tribunaux est un piège pour la justice de proximité et renforcera le phénomène de métropolisation. On va vider chaque tribunal de son contentieux et on annoncera dans quelques années, peut-être, que les tribunaux n'ont plus d'utilité. Le Sénat avait veillé à ce que la nouvelle organisation de la première instance préserve le maillage territorial et la proximité de l'institution judiciaire, en s'assurant, par la mise en place de chambres détachées, qu'aucun site judiciaire ne serait fermé, en prévoyant un mécanisme d'encadrement de toute évolution de la carte judiciaire, et en créant une fonction de juge chargé du contentieux de proximité. C'est en effet une justice proche des citoyens, à la disposition des citoyens qu'il faut préserver. Jugeons des hommes et non des dossiers, n'allons pas vers une justice de médiation, une justice sans oralité des débats dans laquelle certains de nos concitoyens ne se reconnaîtront plus. La justice, c'est l'égalité, l'égalité de toutes et tous devant la loi. Elle doit avant tout être humaine et préserver, bien sûr, la paix dans la société. C'est une impérieuse nécessité, aujourd'hui. L'amendement

parmi nous. Il vise à lutter contre une injustice trop souvent dénoncée dans le cadre des procédures de justice, en particulier par les victimes disposant de peu de ressources, et donc éligibles à l'aide juridictionnelle, cela concerne singulièrement les femmes -mais également par les avocates et avocats des parties civiles. Pour un avocat ou une avocate, consacrer du temps à l'aide juridictionnelle peut représenter un risque ou un sacrifice financier. Ce risque est d'autant plus grand lorsque l'AJ est réalisée pour la victime. En effet, l'AJ est plus

en prévoyant un rapport au Parlement sur l'exécution de la présente loi préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, pratique usuelle en matière de loi de programmation comprenant un volet budgétaire. En second lieu, le projet de loi tel qu'il a été adopté par le Sénat prévoit plusieurs mesures en matière d'aide juridictionnelle, auxquelles le Gouvernement s'est d'ailleurs opposé en raison de la réflexion qu'il mène actuellement sur le sujet. Un rapport conjoint de l'Inspection générale de la justice et de l'Inspection générale

M. Raymond Vall. L'article 2 vise à contraindre les parties à recourir davantage à la médiation et à la conciliation pour régler leurs différends, y compris après la saisine d'un juge. Or nous ne disposons pas d'une démonstration claire de l'efficacité de ces procédures dans l'étude d'impact. Au contraire, celle-ci précise que le nombre de tentatives de conciliation judiciaire était faible jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21siècle, dite la tentative de conciliation préalable obligatoire devant le tribunal d'instance. Aujourd'hui, ce nombre augmente du fait de cette obligation, mais non du fait de l'efficacité du dispositif. Par ailleurs, la médiation à un coût, qui risque de pénaliser les justiciables les plus pauvres. L'étude d'impact précise, là encore, que la médiation est payante- sauf la médiation familiale qui est prise en compte par la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF -, puisqu'il s'agit d'une activité libérale, et les tarifs sont libres. Le coût horaire de médiation est alors variable, de 100 euros à plus de 500 euros, même si des forfaits assortis d'un tarif pour chaque heure supplémentaire effectuée sont souvent proposés, de 500 euros à 1 500 euros. Cet amendement a donc pour objectif de supprimer ces dispositions. l'avis de la commission ? Si la commission a supprimé le II de l'article 2, c'est-à-dire l'extension du champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des litiges préalable à la saisine du juge, elle a en revanche souhaité conserver le I de cet article relatif à l'extension du pouvoir du juge d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, et à la possibilité pour le juge d'ordonner une médiation dans une décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. L'avis est donc défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? l'avis du Gouvernement ? Je rappelle que l'objectif poursuivi par le Gouvernement est le développement des modes alternatifs de règlement des différends pour favoriser l'émergence d'une solution qui ne soit pas nécessairement contentieuse, et ce à tous les stades de la procédure, un accord entre les parties étant susceptible d'intervenir. C'est pourquoi je soutiens l'extension de la tentative obligatoire de résolution amiable des différends préalablement à l'instance, afin que seules les affaires contentieuses qui ont été « décantées » puissent être portées devant le juge. C'était l'objet du II de l'article 2 que votre commission a supprimé. Il est également prévu qu'au cours de l'instance, en tout état de la procédure, le juge pourra enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Enfin, pour permettre une meilleure exécution des décisions en matière d'autorité parentale, le juge pourra ordonner aux parties, dans la décision qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de rencontrer était l'objet de la disposition que le Gouvernement avait proposée. Je rappelle qu'il ne s'agit que d'une possibilité pour le juge. Ce dernier ne pourra enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur que, ainsi que cela est précisé au 2°, lorsqu'il estime qu'une solution amiable du litige est possible. Il me semble qu'il est particulièrement opportun de prévoir cette possibilité,

je parle au nom de Laurence Rossignol. Le règlement amiable des conflits existe en droit de la famille. Cependant, en cas de violences conjugales, le recours à la médiation n'est possible qu'avec l'accord de la victime. Ce principe n'écarte pas un risque majeur pouvant amener la victime à ne pas faire valoir ses droits : il s'agit des cas dans lesquels la victime se trouve dans une situation d'emprise, ce qui pourrait l'empêcher de refuser le recours à la médiation. Le présent amendement vise à maintenir la force de ce principe en le précisant directement dans les articles organisant la médiation dans le cadre des tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps.

son rapport intitulé, la délégation aux droits des femmes du Sénat avait proposé diverses recommandations visant à mieux protéger les femmes victimes de violences. Les rapporteurs Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde,

puisque la commission a supprimé le 1° du I de l'article 2, c'est-à-dire qu'elle a rétabli l'interdiction générale faite au juge de désigner un médiateur pour procéder aux tentatives de conciliation obligatoires prévues en matière de divorce et de séparation de corps, par coordination avec la suppression de l'article 12.

Il va de soi que lorsque le juge est informé de violences intrafamiliales, il ne va pas proposer de médiation aux parties. Il me semble qu'il est important de faire confiance aux juges, qui sont particulièrement sensibilisés sur ces questions. Par ailleurs, je souligne que la nouvelle procédure de divorce prend en compte le dispositif de l'ordonnance de protection, qui est extrêmement utile et permet d'engager une mise en sécurité réelle pour les victimes de violences.

des litiges. C'est un moindre mal, mais cette mesure ne s'oppose pas frontalement à une mesure forte de déjudiciarisation. Comme cela a été dit lors de la table ronde organisée par de nombreux représentants des corps et professions, cette dématérialisation de la justice met en danger la notion même de justice. L'article 3 transfère en effet à des sociétés de droit privé, en quelque sorte, le pouvoir de rendre justice. On voit bien le but de la manoeuvre : désengorger les tribunaux et alléger les coûts. Mais je crois que cela va bien au-delà. Nous avions d'ailleurs contesté en première lecture l'instauration d'une obligation de consultation, car nous estimions qu'elle induisait une forme de privatisation de la justice. Nous y sommes avec cet article 3. De plus, ces dispositions sont source d'inégalités : ces services auront un coût, les start-up du « nouveau monde » sauront en tirer profit, et les plus riches seront bien sûr les mieux servis. Outre la question du coût immédiat de ces services, se pose la question de la fracture numérique. N'oublions pas que plus de 20 % de nos compatriotes sont encore exclus d'internet. Cette mesure est donc grave.

à la démarche gouvernementale. C'est pourquoi nous proposons la suppression de l'article 3. Quel ? Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a considéré en première lecture qu'il était nécessaire d'encadrer les nouveaux services en ligne d'aide au règlement nouveaux services en ligne d'aide au règlement amiable des litiges et d'aide à la saisine des juridictions. Ces services existent déjà il s'agit de les encadrer pour améliorer les garanties pour les justiciables. Supprimer cet article aboutirait à accepter l'absence de toute régulation, ce qui est sans doute contraire aux intentions des auteurs de l'amendement. L'avis est donc défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Comme vient Quel est l'avis du Gouvernement ? Comme vient de le préciser M. le rapporteur, on ne peut pas nier aujourd'hui que ces services en ligne existent. La volonté du Gouvernement est de les réguler

une justice coûteuse et rapide pour les uns, et une seconde lente avec prise en charge par l'aide juridictionnelle pour les autres. La médiation telle qu'envisagée par la réforme risque de retarder

les avocats appliquant d'ores et déjà la règle suivant laquelle « il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès ». Il est clair que cette réforme répond à des préoccupations surtout budgétaires. Si le but est de déjudiciariser, ce délestage ne peut et ne doit pas se faire sans mise en place de garde-fous et sans contrôle de ces sociétés privées. Il ne faudrait pas que, la médiation,

le risque accru d'une justice à deux vitesses. Il risque d'y avoir, à terme, une justice coûteuse et rapide pour les uns, et une seconde La médiation telle qu'envisagée par la réforme risque de retarder et de limiter l'accès au juge et de décourager les justiciables de saisir la justice.

que l'article 226-13 du code pénal est applicable aux personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement de services en ligne de résolution amiable des litiges, toute atteinte au secret professionnel de la part

n° 14 rectifié : la commission a prévu une certification obligatoire de ces services en ligne afin qu'ils puissent être proposés au public, tout en indiquant que les modalités des procédures de délivrance et de retrait de la certification devront être précisées par un décret en Conseil d'État.

l'amendement n° 42. L'article 5 confie aux notaires l'établissement des actes de notoriété constatant la possession d'état en matière de filiation, l'établissement des actes de notoriété suppléant les actes d'état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu à la suite d'un sinistre ou de faits de guerre, ainsi que le recueil du consentement en matière d'assistance médicale à la procréation. En première lecture, le Sénat proposait d'exclure la

nécessitent indubitablement un contrôle du juge, lequel est déjà doté du pouvoir d'appréciation et d'une expérience en la matière. Nous considérons, par ailleurs, que l'ensemble de ces actes doit demeurer gratuit, conformément au principe de service public. Le recours à un notaire se traduira inévitablement par un surcoût pour le justiciable. En outre, nous estimons que cet article, en l'état, constitue un recul intolérable de la protection judiciaire des enfants et des intérêts du plus faible, ce qui risque d'entraîner une fragilisation du droit de la famille. Enfin, mes votre attention sur le fait qu'en outre-mer, et notamment à la Martinique, ces mesures seraient particulièrement dangereuses en raison de très nombreuses difficultés de règlement des successions. C'est pourquoi nous souhaitons la suppression de l'article 5

tels que les actes de notoriété constatant la possession d'état en matière de filiation ou les actes de notoriété qui suppléent les actes d'état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par suite d'un sinistre ou de faits de guerre. Le Gouvernement a étendu le dispositif en confiant au seul notaire le recueil du consentement du couple ayant recours à une procréation médicalement assistée nécessitant l'intervention d'un tiers donneur.

L'efficacité et la force de la justice, en l'occurrence, exigent de conserver la compétence publique. Quel

la possession d'état en matière de filiation et des actes de notoriété suppléant les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par suite d'un sinistre ou de faits de guerre. La commission a estimé que ces transferts s'inscrivaient dans une logique d'uniformisation des règles de compétences applicables à la délivrance des actes de notoriété. Le code civil prévoit en effet deux autres hypothèses dans lesquelles des actes de notoriété peuvent être délivrés : la preuve de la qualité d'héritier et l'hypothèse dans laquelle il est impossible pour l'un des deux futurs époux de fournir un extrait de son acte de naissance avec indication de la filiation. Dans ces deux hypothèses, ces actes sont déjà délivrés par les notaires.

le Sénat en première lecture. Pour rappel, la commission des lois a supprimé l'allégement le plus contestable, qui concernait les actes du tuteur réalisés en matière financière sans contrôle. Elle a par ailleurs refusé de reprendre à son compte toutes les dispositions nouvelles introduites par l'Assemblée nationale en première lecture tendant à accroître le nombre des actes que le tuteur pourrait effectuer seul, sans autorisation préalable du juge. Seraient concernées toutes sortes de décisions : les actes médicaux les plus graves, la gestion des comptes bancaires ou encore la souscription d'une convention obsèques- vos rapporteurs estiment que de telles dispositions porteraient gravement atteinte aux intérêts des personnes

que cet article 8 traduit le premier des deux volets de la grande réforme des tutelles dont il parlait à l'instant. En effet, nous avons reçu un rapport, qui a été rédigé par Mme Anne Caron-Déglise, sur cette question des tutelles. Dans ce rapport figuraient plusieurs recommandations.

Nous avions dit que cette suppression revenait à supprimer le moment où le juge rencontre les époux pour négocier avec eux, discuter et décider des mesures provisoires.

dans la procédure de divorce, c'est-à-dire l'obligation, pour l'époux qui veut divorcer, de solliciter l'autorisation d'introduire la demande et de respecter, ensuite, un délai de réflexion de trois mois avant de pouvoir assigner l'autre conjoint en divorce- tout cela me semble franchement justifié. Dans la rédaction nouvelle issue de l'Assemblée nationale, à l'alinéa 28 de l'article 12, vous prévoyez, ce qui me paraît satisfaisant, que le juge aux affaires familiales doit immédiatement procéder à une audience pour fixer les mesures provisoires.

puisque nous sommes dans la période de représentation obligatoire. Or il est essentiel que, à un moment ou à un autre, les époux qui divorcent puissent rencontrer le juge : il est fondamental que les époux souhaitant divorcer puissent discuter non seulement des pensions alimentaires mais surtout de la résidence des enfants et des modalités de garde.

? Notre collègue a subodoré l'avis de la commission. Cet amendement vise à rétablir l'article 12 supprimé par la commission. Ses auteurs estiment que, dès lors que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale prévoit que le juge tient, dès le début de la procédure, une audience pour fixer les mesures provisoires nécessaires à assurer l'existence des époux et des enfants, la phase de tentative de conciliation ne serait plus nécessaire. Or la commission a considéré que la suppression de la phase de conciliation risquerait de favoriser une logique d'affrontement des parties et, par là même, d'entraîner une augmentation du nombre de divorces pour faute, car la phase de conciliation est une phase de réflexion et de maturation du divorce. Elle a estimé que le problème de la lenteur de la procédure de divorce ne résultait pas tant de la phase de conciliation que de l'insuffisance des moyens octroyés aux juridictions pour se prononcer dans des délais raisonnables. Par ailleurs, si la nouvelle rédaction proposée par l'Assemblée nationale prévoit bien une audience au cours de laquelle le JAF fixe les mesures provisoires, le texte prévoit également que « les parties ou la partie seule constituée » peuvent renoncer à cette audience. En cas de relations houleuses entre les époux, et notamment si une seule des parties est constituée, cette audience pourrait donc ne pas avoir lieu. Cette disposition est par conséquent susceptible de placer l'intérêt supérieur de l'enfant entre les mains de parents qui se déchirent. Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable

Il me semble que l'article 12, qui traite de l'évolution de la procédure du divorce contentieux, est le témoignage parfait d'un travail fait d'écoute

d'une procédure exclusivement écrite pour juger certains litiges dès lors que les parties seraient en accord. Ceux-ci pourraient alors être jugés sans audience. Le règlement des litiges inférieurs à un certain montant, qui sera donc fixé par décret, se ferait également sans audience par le biais de la procédure dématérialisée. dématérialisée. Ces nouvelles mesures portent gravement atteinte au droit des justiciables à un procès équitable et à notre modèle juridictionnel tout entier. Leur seul motif est d'ordre économique et ne saurait justifier les conséquences déplorables qui s'ensuivront. Quel est l'avis de la commission ? Ma chère

constitution d'une instance juridictionnelle nationale qui sera saisie de tous les problèmes d'injonction : cinq magistrats et une vingtaine de greffiers traiteront les 500 000 procédures annuelles

c'est un autre problème : il faut aller vite ; il faut être compétitif ! Vous pensez bien que nous ne saurions accepter ce type de justice automatique. Ce n'est plus de la justice, c'est de la régulation de flux, pour désencombrer les juridictions et faire des économies.

à l'assignation, et afin d'obtenir une décision de justice enjoignant au débiteur de verser les sommes dues. Cette procédure se déroule sans audience : concrètement, le créancier adresse un dossier au juge, qui apprécie le bien-fondé de la demande. Si le débiteur conteste la décision dans le mois suivant la signification de l'ordonnance par un huissier de justice, les parties sont convoquées devant le juge pour un débat dit contradictoire. Il y a chaque année 470 000 requêtes en injonction de payer. Cet article, en instaurant une seule juridiction pour tout le territoire s'agissant des injonctions de payer, pose un problème en termes d'accès au juge. Cet accès sera rendu plus difficile et plus complexe,

dans un tribunal unique, avec des magistrats. Il va de soi que les justiciables pourront saisir la juridiction nationale des injonctions de payer en déposant leur requête, y compris par voie papier auprès du tribunal de proximité, qui la transmettra à la juridiction nationale des injonctions de payer.

alors la vérification exacte des pièces ? Certes, elle aura lieu dans un second temps, si le débiteur prend la précaution de faire opposition à l'injonction de payer. Or il s'agit souvent de débiteurs impécunieux et peu avertis des règles de droit.

de la procédure d'injonction de payer. Lorsque la requête aux fins d'injonction de payer est déposée, le débiteur n'est pas au courant-

inexact- sans doute n'a-t-il pas une connaissance très précise de ce sujet. Il est écrit que « cet accès sera rendu plus difficile et plus complexe car les justiciables devront former opposition devant la juridiction unique nationale et donc se déplacer jusqu'à cette juridiction pour assister à l'audience ».

Cet amendement a deux objets. D'une part, il s'agit de rendre possible la dématérialisation de « l'opposition aux demandes d'injonction de payer » et non pas seulement la dématérialisation des des « demandes d'injonction de payer », comme le prévoit l'article dans la rédaction issue de l'examen en commission. D'autre part, il s'agit de revenir sur la suppression des audiences pour le traitement des oppositions aux demandes d'injonction de payer, lorsque l'opposition tend exclusivement à l'obtention de délais de paiement. Beaucoup de justiciables poursuivis par des organismes de crédit ou des bailleurs ont déjà du mal à exprimer oralement leur prétention, qu'en sera-t-il lorsqu'ils devront le faire exclusivement par écrit, par le biais d'une plateforme numérique ? En l'état, cette disposition est susceptible de porter atteinte au principe du contradictoire, notamment au regard du taux d'illettrisme de certains départements, tels que la Martinique, où ce taux est près de six fois supérieur à celui de l'Hexagone. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement de la commission ? Cet amendement tend à modifier la procédure relative aux oppositions aux injonctions de payer pour prévoir qu'elle peut se faire par voie dématérialisée et supprimer la possibilité de traitement de ces dossiers sans audience devant le juge. Or l'article 13 prévoit que les oppositions aux injonctions de payer en deçà d'un certain montant pourront se faire par voie dématérialisée, si les parties en sont expressément d'accord.

Cet amendement vise à supprimer la notion de recours aux forces de police pour faire exécuter les décisions des juges aux affaires familiales, au regard des dérives d'ores et déjà constatées du point de vue de l'utilisation du syndrome d'aliénation parentale pour faire peser sur les mères une présomption de culpabilité. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement est contraire à la position de la commission. Il tend en effet à supprimer tous les outils prévus à l'article 18 pour améliorer l'exécution des décisions prises en matière l'autorité parentale. L'objectif de cet article est d'apporter une réponse graduée à ces inexécutions, allant de la médiation familiale jusqu'à la réquisition des forces de l'ordre pour les hypothèses les plus graves. L'avis est par conséquent défavorable

de magistrat. Nous partageons l'avis des professionnels qui considèrent que cette possibilité serait « symboliquement désastreuse pour des magistrats par nature très expérimentés qui se trouveraient ainsi, dans le cadre de l'honorariat, dans une situation d'infériorité par rapport à leurs collègues en activité ». L'objectif est clair pour le Gouvernement mais aussi pour la majorité sénatoriale qui accepte cette qui accepte cette disposition : faire des économies. Faire partager l'expérience des plus anciens est une bonne chose, mais cela ne doit pas se substituer au recrutement de nouveaux magistrats, dans une justice administrative qui est sous grande pression. À nos yeux, cette disposition est un pis-aller et nous ne l'acceptons pas. nous ne l'acceptons pas. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour des magistrats honoraires d'assurer des fonctions d'aide à la décision auprès d'autres magistrats. Or cette possibilité est déjà prévue pour les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire à l'article 40 de la loi organique du 8 août 2016. Par ailleurs, la commission a précisé, comme à l'article 40, que ce n'est qu'à leur demande que les magistrats honoraires des juridictions administratives pourront être désignés pour assurer ces fonctions. Par conséquent, l'avis est avis défavorable

84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, « tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics ». L'étude d'impact établit le nombre de magistrats Le recours à ces magistrats a progressivement été étendu à partir de 2006, d'abord pour les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière. Le CESEDA, ou code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permet qu'ils statuent seuls sur les recours formés par les demandeurs d'asile placés en rétention ou qu'ils soient rattachés à certaines juridictions spécialisées, comme la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Cette faculté a par ailleurs été considérablement ouverte dans l'ordre judiciaire

le recours à ces magistrats dans l'ordre administratif. En parallèle, les règles de déontologie s'imposant aux magistrats honoraires voulant exercer comme avocat relèvent du « droit mou » de la charte de déontologie de la juridiction administrative du 14 mars 2017. Compte tenu des nouvelles fonctions juridictionnelles qu'il est prévu de leur confier et qui leur permettront de « garder un pied » dans les juridictions, il convient de prévenir au maximum les risques de conflits d'intérêts pouvant survenir à cette occasion, en étendant l'encadrement du cumul d'activité juridique et judiciaire en France et à l'étranger. En effet, il n'est pas rare que d'anciens magistrats administratifs ou membres du Conseil d'État soient recrutés par des cabinets étrangers. Quel est l'avis de la commission

à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d'être salariés d'un membre d'une telle profession, ou d'effectuer un acte d'une telle profession à l'étranger. L'article 18 ne prévoit de telles incompatibilités qu'en France. Cela nous paraît suffisant, d'autant qu'une telle interdiction pour des activités menées à l'étranger ne nous semble pas exister pour les magistrats administratifs en fonction ou pour les magistrats judiciaires en fonction ou honoraires.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement vise à garantir le maintien de l'oralité lors de la révélation des faits de violences à caractère sexuel. Cette oralité est indispensable pour poursuivre le mouvement de libération de la parole des victimes, mais également parce que les témoignages de vive voix, dans la mesure du possible filmés, constituent des éléments de preuve cruciaux dans le cadre de la procédure d'instruction, puis du jugement.

rectifié. Il s'agit de garantir aux victimes d'infractions sexuelles le droit à l'intimité lorsqu'elles viennent témoigner de l'agression subie. En effet, les témoignages de victimes ayant souffert d'avoir dénoncé leur agression en présence de tiers, voire à l'accueil du commissariat ou de la gendarmerie sont nombreux. Ce traumatisme s'ajoute à celui qu'elles ont subi lors de l'agression sexuelle ou du viol, nuit au processus de reconstruction des victimes et crée chez elles un fort sentiment d'injustice. Cet amendement vise donc à permettre aux victimes de témoigner dans un lieu apte à recevoir leur parole.

Le fait d'inscrire dans la loi que l'intimité de la personne doit être respectée dans les conditions dans lesquelles elle est accueillie

sera un argument dans un certain nombre de situations et une incitation à faire en sorte qu'il y ait une salle, un lieu où l'intimité puisse être respectée. Il me paraîtrait assez

permettra de faire avancer les choses et poussera le Gouvernement- s'il en a les moyens, j'espère qu'il le fera -à améliorer les locaux des commissariats. Pour ma part, je voterai cet amendement.

elle-même. Or c'est déjà si difficile et si compliqué de venir déposer plainte ! Une fois amendé, cet article renforcera le droit au dépôt de plainte, en prévoyant que, sauf refus express de la victime, la prise de plainte est obligatoire lors de la dénonciation d'infractions à caractère sexuel. L'amendement

Gouvernement ? Même avis. Si une difficulté ponctuelle surgit- nous ne nions pas que cela puisse arriver -, la procédure consiste à écrire au procureur de la République, qui demande immédiatement au commissaire de police de prendre en charge cette plainte.

Je vous remercie,

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent une intrusion sans commune mesure dans la vie privée du justiciable. Les mesures qu'elles permettent, extrêmement attentatoires au respect de la vie privée, sont autorisées avec beaucoup de précautions et ont commencé à être encadrées en France par la loi du 28 mars 2014. Cette ingérence généralisée ne semble pas poursuivre un but nécessaire et légitime. Par ailleurs, l'article prévoit une nette extension ce qui fait craindre un cruel manque d'indépendance dans la tenue des enquêtes et la disparition,, du juge d'instruction. En effet, on observe une extension inquiétante des pouvoirs du parquet et des officiers de police judiciaire, les pouvoirs initialement dévolus au juge d'instruction étant étendus au procureur de la République. Un tel article ne saurait être accepté ni même amendé. Certains ont proposé de porter le seuil de trois ans à cinq ans pour que ces mesures ne s'appliquent légalement qu'aux crimes et délits punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, au nom du principe de précaution, eu égard aux risques de dérives sécuritaires, nous demandons la suppression pure et simple de cet article.

et portent gravement atteinte aux libertés publiques. Nous regrettons que la navette parlementaire n'ait pas permis d'avancer sur ce point. La majorité sénatoriale, pourtant consciente des menaces potentielles contre les libertés individuelles, s'est obstinée dans la recherche d'un hypothétique compromis, lequel ne viendra pas. Cet article étend le recours à la géolocalisation et aux interceptions par voie de communications électroniques aux enquêtes préliminaires et de flagrance pour les crimes et délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Alors que l'opinion et les juristes s'inquiètent

Voter ces amendements, c'est supprimer ces dispositifs. La commission des lois n'a pas fait ces choix-là. Elle maintient ces dispositifs, considérant qu'ils ont leur utilité. Elle les a simplement encadrés,

? Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces amendements. Je rappelle que les mesures que nous proposons résultent des propositions formulées dans le cadre des chantiers de la justice, qui ont eu lieu l'année dernière. Au fond, nous avons voulu simplifier et rapprocher les régimes les régimes d'utilisation de ces interceptions téléphoniques ou de la géolocalisation. Il me semble en effet que rien ne justifie que les interceptions téléphoniques ne soient actuellement autorisées au cours d'une enquête que pour des faits de délinquance ou de criminalité organisée alors alors qu'elles sont très largement possibles à l'instruction pour toute infraction punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement. Cette différence de champs d'application, selon le type de procédure, qu'il s'agisse de l'enquête ou de l'instruction, est propre aux écoutes et n'existe pas pour les autres mesures. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité procéder à une simplification. En outre, les garanties qui sont prévues lors de l'enquête sont équivalentes à celles de l'instruction dès lors que, dans les deux cas, elles seront autorisées par un magistrat du siège, soit le juge d'instruction, soit le juge des libertés et de la détention. Enfin, il nous semble que la seule différence qui soit justifiée, et qui demeure dans notre texte, c'est la durée

un contrôle du juge des libertés et de la détention, l'obligation de motivation d'usage des écoutes téléphoniques par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, l'amélioration du contrôle, ainsi que les limites du recours à la géolocalisation. Toutefois, il faut être bien conscient que ces techniques sont très intrusives. Elles portent nécessairement atteinte à la vie privée. On peut comprendre que les enquêteurs aient envie de ne pas en être privés dans le cadre

En première lecture, le Sénat avait effectivement retenu le seuil de trois ans d'emprisonnement, et non de cinq ans, comme le proposent les auteurs de l'amendement, afin que les techniques de géolocalisation puissent être utilisées dans le cadre d'affaires d'évasion. Je parle bien d'évasions. Il nous semble en effet utile que la géolocalisation puisse être utilisée en pareille circonstance. Nous avions également considéré que cette technique n'impliquait pas le même degré d'intrusion dans la vie privée que d'autres techniques d'enquête et que le seuil de trois ans était, de ce fait, parfaitement acceptable. En contrepartie, nous avions demandé que l'autorisation de recourir à la géolocalisation soit motivée et renouvelée tous les quinze jours, et non tous les mois,

l'amendement n° 18 rectifié. Cet article prévoit la généralisation de l'enquête sous pseudonyme à l'ensemble des crimes et délits passibles d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. Il étend la possibilité pour les cyberpatrouilles de réaliser des enquêtes sous pseudonyme. Dans le texte initialement présenté par le Gouvernement, ces enquêtes devaient être ouvertes pour tous les crimes et délits. La condition des trois ans d'emprisonnement, introduite lors des travaux au Sénat, vient un peu limiter sa portée, qui avait été jugée trop large.

de telles mesures pour l'ensemble des infractions pénales, et celles qui sont punies de trois ans d'emprisonnement, sont évidentes. Le contrôle par l'autorité judiciaire n'est pas suffisant, d'autant que c'est une fois encore sous l'autorité du procureur de la République que s'effectueraient de tels actes.

l'amendement n° 52. L'article 28 vise à étendre le recours et l'enquête sous pseudonyme aux cyberinfiltrations. Ce dispositif existe déjà dans le droit pénal français, est pour le moment limité aux enquêtes en matière de criminalité et de délinquance organisée, soit pour des méfaits extrêmement graves, ce qui classe cette mesure dans le régime d'exception. L'article initial du projet de loi était excessif, car il visait à généraliser cette mesure à toutes les enquêtes liées à un délit ou un crime entraînant une peine d'emprisonnement. Cette extension paraissait dangereuse dans la mesure où elle mettait fin au monopole de l'emploi de cette mesure par des services spécialisés. Or une telle technique d'enquête, équivalant à l'infiltration, ne peut être efficace que si elle est mise en oeuvre par des personnels spécialement formés à la spécificité de la cybercriminalité, et plus particulièrement aux techniques d'infiltration numérique. La commission des lois a assoupli le dispositif prévu dans le texte au travers d'un amendement du rapporteur visant à cantonner l'extension de cette mesure aux infractions punies d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement. Elle a également accru le contrôle des magistrats lorsqu'une enquête sous pseudonyme sera diligentée. Mes chers collègues, nous notons évidemment les améliorations et apports venus modifier l'article 28. Nous réprouvons simplement le recours même à ce type d'enquêtes qui portent atteinte au principe de la loyauté de la preuve. Aussi le présent amendement tend-il à supprimer l'article 28. La parole

ailleurs, nous avons souhaité, contrairement à ce que j'ai entendu, renforcer le contrôle de l'autorité judiciaire : nous exigeons l'autorisation préalable d'un magistrat lorsqu'il y a acquisition ou transmission de produits illicites,

ait restreint le champ de l'enquête sous pseudonyme aux seules infractions punies d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement. J'avais eu l'occasion de le dire en première lecture, il nous semble que cela constitue un recul

explication de vote. À titre personnel, je ne voterai pas ces amendements de suppression, car je pense qu'il faut trouver de bons compromis. Il s'agit ici de permettre à la police de mener des enquêtes sous pseudonyme, notamment dans les communications électroniques. On sait très bien quel est l'enjeu aujourd'hui : il s'agit de pouvoir traquer un certain nombre d'acteurs qui commettent des infractions ou qui provoquent à la commission d'infractions par ce biais-là. Vous avez proposé, messieurs les rapporteurs, que le recours à cette mesure soit limité à des infractions sanctionnées de peines d'emprisonnement de trois ans. Mme la ministre dit que cela ne couvre peut-être pas tous les champs ; dans ce cas, il faudrait les préciser. Il est vrai que ce sont des sujets extrêmement délicats.

est-il illusoire, mais conservons-le jusqu'à la fin de nos débats -étant de convaincre les collègues députés à l'Assemblée nationale qu'il y a du bon dans le texte du Sénat et qu'ils doivent en reprendre certains éléments. Prenons peut-être ce chemin-là sur cet article-là.

Mme la garde des sceaux. C'est un amendement de coordination. Le nouvel article 230-46 du code de procédure pénale, relatif à l'enquête sous pseudonyme, prévoit que les officiers de police judiciaire doivent, pour procéder à de telles enquêtes, être spécialement habilités, dans des conditions déterminées dans un texte réglementaire. Les officiers des douanes judiciaires, qui sont affectés dans le service national de douane judiciaire, disposent des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire. Il apparaît également nécessaire de déterminer

Merci